Nous reprenons la séance. Et la parole est d'abord à Madame. Esther Benbassa, pour une mise au point. Sur un vote. écrit le président. Je souhaite faire une mise au point sur le scrutin numéro 124. J'aurais souhaité voter pour.

Didier Rambaud a souhaité voter pour et Alain Richard n'a pas souhaité prendre part au vote. Je vous remercie. Merci madame. Ah les données de ces mises au point et elles seront publiés au JO et figureront dans l'analyse politique. Maintenant monsieur Folliot à la parole pour un rappel au règlement. Merci monsieur le président. j'ai pas pu faire l'explication de vote et en deux mots, c'est dire que moi je soutiens bien sûr tout à fait le travail de mémoire qui est fait par rapport à ce qui est réellement un génocide et que j'ai pris une position depuis quelques années qui était de refuser de voter les lois mémorielles. C'est-à-dire qu'en fait je suis tout à fait d'accord sur le, sur le principe mais par rapport aux éléments mais que je trouve dangereux et ce que je mette expliqué Hans là en commission de la Défense et des Affaires étrangères pour dire que je trouvais que voter des lois mémorielles était un engrenage dans lequel nous étions et qui parfois pourrait nous mettre dans des situations un peu difficile. Voilà, merci. Voilà que données de votre rappel au règlement. Mes chers collègues les connus les conclusions adoptées tout à l'heure. Pendant, pendant ce même débat par la conférence des présidents réunie ce jour 100 consultable sur le site du Sénat. En l'absence d'observation. Je considère ces conclusions comme adopté. L'ordre du jour à présent. Appelle la discussion de la proposition de résolution européenne. En application de l'article 73 qui inquiète de notre règlement. Sur l'avenir de l'Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes mieux connu sous le nom de Frontex résolution présentée par le président Rapin hein et le président François-Noël Buffet. C'est une demande du groupe S E R et du groupe écologiste. Dans la discussion générale la parole d'abord au président Jean-François Rapin. Pour cinq minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, cher François Noël. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Notre débat en séance publique sur l'avenir de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de gardes-côtes et bienvenue. En effet, le gouvernement présente un nouveau projet de loi immigration en particulier pour réformer le régime de l'asile et pour régulariser les travailleurs sans papiers présents sur notre territoire. notre politique migratoire, mais aussi notre politique de l'asile et de contrôle de nos frontières relève aujourd'hui de compétences partagées avec l'Union européenne. De fait, ces politiques se jouent aujourd'hui en grande partie aux frontières extérieures de l'Union européenne car l'existence de l'espace Schengen. Espace libre de circulation dans tous nos concitoyens profit pour étudier travailler ou voyager dépend d'une surveillance efficace de ses frontières extérieures. Cette mission de gestion et de surveillance des frontières extérieures relève en 1er lieu des États. Mais pour cela, ils peuvent faire appel au soutien opérationnel de Frontex. Cette agence incarne alors la solidarité européenne en déployant des agents et des équipements pour le contrôle des voyageurs aux frontières ou la lutte contre l'immigration irrégulière. La France elle-même bénéficie de cet appui, par exemple sur la Côte d'Opale dont je suis originaire pour surveiller les embarcations de migrants essayant de traverser la Manche vers le Royaume-Uni ou organiser des opérations de retour des migrants irréguliers. Dans leur pays d'origine. Frontex dispose à cet égard des moyens nécessaires pour assurer ce soutien. Elle est dotée cette année d'un budget de 845 millions d'euros et emploie environ 2000 personnes. Ce nombre devant progressivement augmenter pour constituer un contingent permanent de 10.000 officiers en 2027. Mais l'agence Frontex a été paralysé pendant de trop longs mois par une double crise, cette crise a d'abord été la crise de croissance, d'une agence dotée de moyens importants à compter de 2019, mais qui n'a pas eu le temps de procéder aux recrutements nécessaires et de mettre en place de procédures d'audits et de contrôles suffisante. Cette crise a également été une crise de confiance lorsque l'agence a été accusé de manquement dans son fonctionnement interne mais aussi de complicité de refoulements illégaux de migrants en mer Égée en particulier l'agence à leur fait l'objet d'un nombre inédit d'audits et d'enquêtes qui ont conduit à la démission de son ancien directeur Fabrice et Jerry en avril dernier puis à une longue phase transitoire de huit mois enfin terminé le 20 décembre dernier avec la désignation d'un nouveau directeur, le Néerlandais Hans Liechtens qui nous l'espérons ouvre une nouvelle ère. Il est en effet urgent de réagir. 330.000 francs franchissement irrégulier des frontières extérieures de l'Union européenne ont été recensés en 2022, soit une hausse de 64% par rapport à 2021 et une augmentation inédite depuis 2016, Frontex doit se remettre très vite au travail. Il en va de la crédibilité de l'Union européenne et de l'avenir de l'espace Schengen. C'est l'objet de la proposition de résolution européenne que le président Buffet et moi-même avons déposé. Nous avons souhaité par ce texte formulé plusieurs recommandations simples pour que l'action de Frontex représente une valeur ajoutée et non une source supplémentaire de complexité, voire de contentieux. Je veux d'ailleurs remercier nos collègues rapporteur Arnaud de Belenet et Claude Kern qui ont souhaité préserver la cohérence de notre dispositif. J'insisterai sur 3 points. D'abord l'agence Frontex doit exercer sa mission, à savoir soutenir les États membres dans la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne en respectant les droits fondamentaux naturellement mais sans pour autant se transformer en agence de droits fondamentaux ou en agence de l'asile. En effet, ces structures existent déjà au niveau européen ensuite. Frontex n'a pas vocation à remplacer les services douaniers et policiers des États. Mais pour agir en totale complémentarité avec ces derniers. Elle doit faire l'objet d'un pilotage politique plus musclée par le ministre de l'intérieur des États à qui il revient de lui fixer des priorités claires ce pilotage politique doit aussi passer par un suivi et un contrôle de Frontex par le Parlement européen et par les parlements nationaux. Il s'agit d'un enjeu démocratique et d'une demande récurrente de notre commission des Affaires européennes sur laquelle je pense. Nous pouvons tous nous retrouver. Nous autres parlementaires nationaux sommes plus au fait des attentes de nos concitoyens et nous devons donc prendre toute notre part de ce contrôle, pour obtenir des résultats concrets sinon les États se détourneront de Frontex. Je vous remercie. Merci monsieur le président et la parole est ensuite. Le président buffet, coauteur de la proposition de résolution également pour cinq minutes puisque. L'auteur bénéficie de 10 minutes et qu'elles ont été partagées. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur rapporteur chers collègues comme l'a rappelé le président Rapin Frontex se trouve aujourd'hui à un moment critique de son histoire, son action est remise en cause de toutes parts, pourtant elle n'a jamais été aussi capital. Le retour des flux d'immigration irrégulière important la tentative d'instrumentalisation de ces flux par la Biélorussie à l'Automne 2021 ou le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a un an sont autant d'exemples démontrant la nécessité d'une agence en pleine possession de ses capacités. Dans ce contexte, il nous incombe en tant que parlementaires nationaux de faire entendre notre voix pour soutenir Frontex. Il est plus que temps que l'Agence surmonte cette période de turbulences pour se consacrer pleinement et exclusivement à sa mission de gestion des frontières. Avec Jean-François Rapin. Nous avons tenu à ce que la proposition de résolution débute par l'expression d'un soutien clair et sans ambiguïté à cette agence. C'est là le coeur de notre démarche. L'espace Schengen et l'un des acquis les plus précieux de la construction européenne, mais la fin des frontières intérieures n'a de sens que dans la mesure où nous maîtrisons collectivement nos frontières extérieures, l'action de la France est à cet égard absolument décisive. Je rappelle que l'Agence déploie actuellement plus de 2150 hommes et femmes sur le terrain, 10 avions et 22 bateaux en appui des États membres les échanges que j'ai pu avoir avec une délégation de la commission des lois avec la direction de Frontex à Varsovie en avril 2022, n'ont fait que renforcer ma conviction que l'élargissement du mandat de l'Agence va dans le bon sens et qu'il faut la soutenir dans sa mise en oeuvre en conséquence la proposition de résolution européenne que nous présentons ce soir. Salut le choix fait par le législateur européen en 2019. 2 transformer Frontex en une véritable entité opérationnelle avec une capacité de projection autonome la multiplication par 10 de son budget en 10 ans et la création d'un contingent permanent de gardes frontières sont des avancées majeures. Pour autant. Notre soutien n'est pas sans conditions. En particulier, vise à celui du respect des droits fondamentaux. Aucune concession ne peut être faite sur ce point. D'aucuns voudraient opposer le contrôle des frontières au respect des droits fondamentaux. Bien évidemment cela n'a pas de sens tant les 2 vont de Pair. Notre soutien à Frontex ne peut ensuite se résumer à des mots. C'est pourquoi notre texte comprend des recommandations recommandations concrètes pour accompagner l'agence vers la sortie de crise. Pour ce faire, il nous paraît d'abord indispensable de mettre en place un vrai pilotage politique de celle-ci. Le nouveau directeur exécutif récemment nommé doit pouvoir bénéficier de lignes directrices forte et claire dans son action. Nous proposons pour cela que des réunions du Conseil de l'Union européenne soit spécifiquement dédiée au pilotage politique de Frontex. Les parlements nationaux ont également toute leur place dans cette démarche. On ne peut que regretter que le Parlement européen et décidé de manière unilatérale de former un groupe de contrôle de Frontex et ce alors que le règlement de 2019 prévoit explicitement et je dis bien explicitement une association des Parlements nationaux. La création d'un groupe de contrôle parlementaire conjoint nous paraît être la voie à suivre, comme cela a déjà été fait avec succès à avec pour l'agence Europol. un point crucial et enfin. Celui du dispositif de protection des droits fondamentaux de Frontex. Le constat est sans appel, les procédures existantes n'étaient pas suffisamment robuste pour prévenir et traiter efficacement les incidents survenus en mer Égée. Les réformes du dispositif de signalement des incidents et du mécanisme de traitement des plaintes mises en place par la direction intérimaire vont, de ce point de vue dans le bon sens, de même que le recrutement de 46 contrôleur aux droits fondamentaux. Nous avons toutefois souhaité émettre plusieurs recommandations afin de prévenir l'émergence d'une guerre des chefs de guerre des chefs entre guillemets naturellement chacun l'aura bien compris au sein de l'agence. Par exemple, avec l'instauration de canaux de dialogue renforcé un examen des décisions de l'officier aux droits fondamentaux par le médiateur européen ou encore l'établissement de critères de recrutement exigeant pour l'officier et les contrôleurs aux droits fondamentaux. Je voudrais avant de terminer ce propos remercier notre collègue Arnaud de Belenet, rapporteur de la commission des lois pour les précisions utiles qu'il a apportées au texte sur ce dernier point enfin, nous avons été voulu exclusivement. Exclure. L'hypothèse d'une révision du mandat de Frontex. La priorité est en effet de sortir l'agence de la crise et du lui accorder le temps nécessaire pour accorder pleinement et intégralement son mandat mais. Merci président. La parole est maintenant. Monsieur Arnaud de Belenet, rapporteur de la commission des lois à 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, messieurs les présidents de commission, chers collègues. La proposition de résolution européenne relative à l'avenir de l'Agence européenne des gardes-frontières et de garde-côtes. Initiée par les présidents de la commission des affaires européennes et des lois. Jean-François Rapin et François-Noël Buffet intervient. Ça vient d'être dit à un moment décisif. L'Agence. Traverse une double crise dans sa jeune histoire. Et elle a besoin aujourd'hui d'être conforté. La première de ces crises est structurelle. Elle trouve ses racines en 2015 lorsque l'Union européenne a échoué à répondre efficacement et de manière coordonnée à la crise migratoire en réaction, Frontex a vu son mandat et ses moyens continuellement et massivement renforcé de révisions successives de son mandat en 2016 et 2019 ont considérablement élargi son Champ de compétences, l'agence n'intervient plus uniquement pour répondre à des situations d'urgence mais également via des déploiements sur le terrain de longue durée. Le périmètre géographique de son intervention ne se limite plus à l'espace Schengen puisqu'elle peut également assisté dans la gestion de leurs frontières des pays tiers ayant conclu un accord avec l'Union européenne. Pour mener à bien ces nouvelles missions Frontex a bénéficié d'une progression inédite dans l'histoire de l'Union et de ses moyens. Son budget a été quasiment multiplié par 10 en 10 ans pour atteindre les 145 millions. Cette année, quant à ses effectifs du contingent permanent de garde-frontières devrait atteindre 10.000 personnels. En 2027, jamais une entité européenne ne s'était vu attribuer de tels moyens de telle prérogative de puissance publique, et encore moins d'agents armés et vêtus d'un uniforme à ses couleurs. Depuis sa création en 2004 en moins de 20 ans. Frontex est devenue l'agence la plus puissante de l'Union européenne. En plein changement de dimension Frontex a été sursollicité est confronté à une. Conjonction de crise internationale. Pour citer. Pour s'il fallait en citer je n'en citerai que de la, la tentative d'instrumentalisation des migrations par la Biélorussie à l'Automne 2021 ou l'agression russe en Ukraine. Frontex éprouvé déjà de grandes difficultés pour mener à bien cette transformation dans les délais impartis. L'agence n'était pas outillé pour conduire une réforme aussi ambitieuse aussi rapidement en matière de ressources humaines ou de passation de marchés publics par exemple. Elle ne disposait pas de service suffisamment robuste pour piloter cette évolution dans de bonnes conditions. La directrice exécutive par intérim de l'agence l'indiquer devant nos commissions cet Automne. Je la cite, la pression politique était forte et les délais extrêmement. En conséquence, la croissance de l'agence a entraîné des difficultés opérationnelles. La seconde crise qu'affronte Frontex relève de la confiance, elle touche au respect des droits fondamentaux et à la réputation de l'agence Frontex a fait l'objet d'accusations par des ONG et des médias d'investigation sur sa participation alléguée à des opérations de refoulements en mer Égée. Des enquêtes. Ont été menées. Par le Parlement européen le médiateur européen et l'Office européen de lutte antifraude elles aboutissent à 3 conclusions. L'agence n'a pas participé directement à des pushback mais informer de potentielles violations des droits fondamentaux par les gardes-côtes elle elle a fait preuve d'une passivité tout à fait anormal. Les dispositifs de traitement et c'est le second. Le la seconde conclusion de ces enquêtes, les dispositifs de traitement des incidents n'étaient pas suffisamment robuste pour traiter de situations aussi problématique. Et en dernier lieu, la direction de Frontex a échoué dans sa gestion managériale et a manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de l'Union. Depuis, l'agence est en proie à une crise profonde et durable. Elle a atteint son apogée en 2022 en avril avec la démission de son directeur exécutif notre compatriote Fabrice Leggeri. Et ce n'est d'ailleurs que tout récemment qu'un successeur, a pu être nommé à l'issue d'un. Long et fastidieux processus de désignation. Cette crise a aussi révélé. Outre des inimitiés personnelles l'existence d'un débat au sein des institutions européennes sur la sur les priorités de l'agence 2 visions s'affrontent, la première est centré sur l'objectif de protection des droits fondamentaux et la seconde sur l'obtention de résultats probants en matière de lutte contre en matière de lutte contre l'émigration Éric l'immigration irrégulière. Dans ce contexte, et alors que se pose la question d'une éventuelle révision du mandat de l'Agence à fin 2023. La proposition de résolution de nos 2 présidents permet au Sénat, un positionnement clair sur. Notamment 2 objectifs. Le 1er politiques. Sur le sens à donner au mandat de Frontex en réalité. Nous en avons convenu en commission le débat opposant contrôle des frontières d'un côté et respect des droits fondamentaux de l'autre et largement monté en épingle la première mission de Frontex et le contrôle des frontières, et elle doit s'en acquitter, dans un respect absolu des droits fondamentaux, ce sont bien évidemment là encore les 2 faces d'une même médaille. Le second. Objectif et juridiques et pratiques. Il concerne l'éventuelle révision du mandat de de Frontex. Cette option est explicitement écarté dans la proposition de résolution afin d'accorder à Frontex. Le temps nécessaire pour assumer pleinement son mandat actuel. Comme la commission des Affaires européennes. La commission des lois et sous réserve pour la commission des Affaires européennes de ce que, de ce qu'exprimera le rapporteur Claude Kern tout à l'heure. La commission des lois souscrit pleinement à ces orientations. Le soutien des parlements nationaux et nécessaire à Frontex, celui du Sénat et formulée par le, par une proposition de résolution très clair. Alors que la pression migratoire aux frontières de l'Union européenne. Renoue avec des niveaux très préoccupant. Il est impératif que Frontex soit pleinement au travail. Je rappelle que les passages clandestins vers l'Europe ont encore augmenté en 2022 de 64% et 250% pour la seule route des Balkans. Mais faut également rappeler que la France s'appuie grandement sur Frontex. Notamment, dont nos arrêts dans dans nos aéroports que ce cette intervention sera encore renforcé cette année. Et sur la Côte d'Opale. Nous avons. Directement intérêt à ce que l'Agence laisse la crise derrière elle pour se concentrer sur l'exercice de ses missions soutenir politiquement Frontex n'est toutefois pas suffisant. Nous devons également être force de proposition. C'est le cas de de ce texte qui veut renforcer le pilotage politique de l'agence, par la mise en place de réunion du Conseil de l'Union. Européenne spécifiquement dédiés à son pilotage ou par le rehaussement durant hiérarchique des membres du conseil d'administration. C'est également. Le cas. Nous sommes également force de proposition. S'agissant du dispositif de protection des droits fondamentaux. La commission des lois est très claire sur ce point. Frontex a besoin d'un officier aux droits fondamentaux indépendant et fort. Ce n'est pas une contrainte juridique. De plus, c'est bien une garantie de crédibilité pour l'institution. Mes chers collègues, la Commission partage les objectifs l'esprit et la lettre de la résolution européenne qui nous est proposé par les présidents buffet et Erap hein. Je vous invite à la soutenir ce soir à votre tour et vous remercie de votre attention. Merci monsieur le rapporteur. Et nous en venons à l'intervention de Claude Kern, rapporteur pour avis de la commission des affaires. Dès qu'il y a cinq minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de conversion gère cher François Noël cher Jean François. Monsieur le rapporteur. Chers Arnaud. Mes chers collègues, je voudrais d'emblée remercier nos présidents Jean-François Rapin et Jean et François Noël Buffet pour leur proposition de résolution européenne. Cette dernière est le fruit de leur longue réflexion sur un sujet qu'ils connaissent bien. Et qui nous préoccupe tous, la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne. Car, comme cela vient d'être rappelé l'enjeu du bon fonctionnement de l'agence européenne de garde-frontières et de gardes-côtes Frontex n'est pas un enjeu technique. Ils concernent notre quotidien. Notre libre-circulation dans l'espace Schengen. Et notre maîtrise de l'immigration. En effet les dysfonctionnements aux frontières extérieures ont des conséquences immédiates avec des mouvements de migrants irréguliers, important vers la France et toutes les conséquences qui en découlent et que nous pouvons constater au niveau local en terme de précarité, de besoin de structures d'accueil et de trafic d'être s'humains. Bien sûr que c'est aux États d'assumer en premier ressort leur leur mission de gestion et de surveillance des frontières, mais ils doivent aussi pouvoir s'appuyer sur une agence Frontex opérationnel et réactive. Comme elle vient de le démontrer, aux frontières de l'Ukraine. Pouvoir s'appuyer sur une agence Frontex respectueuse des droits fondamentaux qui est à même de se retirer d'une opération menée avec un membre. C'est les agents de ce dernier commettre des irrégularités. Pouvoir s'appuyer sur une agence Frontex enfin qui sait où sont ses priorités. Car elle fait l'objet d'un vrai pilotage politique et d'un contrôle associant Parlement européen et Parlements nationaux. Voilà pourquoi lors de sa réunion du 14 décembre dernier. La commission des Affaires européennes a approuvé la proposition de résolution européenne qui fait l'objet de notre discussion de ce soir sans la modifier. Les dispositions du texte demandant contrôle parlementaire conjoint. De l'Agence par le Parlement européen et les parlements nationaux ont d'ailleurs recueilli un consensus. La commission des lois ensuite procéder à son propre examen du texte est adopté 3 amendements qui actualise les dispositions de la résolution. Elle a aussi adopté un amendement de précision utile sur l'expérience requise de l'officier au droit fondant fondamentaux et des contrôleurs aux droits fondamentaux. En effet il semble pertinent que l'officier puisse attester d'une expérience approfondie en matière de gestion des frontières. Quand les contrôleurs devraient pour leur part, prouver une expérience opérationnelle en matière de surveillance des frontières. Ces amendements sont respectueux du souhait des auteurs de la proposition. Et du vote de notre commission, nous y sommes donc favorables. En revanche, je rappelle qu'une proposition de résolution est un voeu politique qui a sa cohérence, tout comme le vote de notre commission. Par conséquent, tout en respectant la vision de chacun je serai défavorable à tous les amendements déposés. Qui dénature son dispositif ou le rendre inopérant. Avec cette proposition de résolution nous adressons en effet un message important aux institutions européennes. Frontex est une belle réalisation européenne. Un projet de coopération concrets et ambitieux mais elle doit encore démontrer sa valeur ajoutée, sans renoncer un instant à notre contrôle démocratique. Il faut laisser travailler Frontex dans la sérénité. Sinon sans son aide précieuse certains États particulièrement exposés exposées à la pression migratoire renonceront à leurs obligations de surveillance et d'enregistrement aux frontières et nous serons de nouveau face à des flux incontrôlé et au au retour de chaque du chacun pour soi. Merci pour votre attention. Monsieur le président. C'est le président de la commission des lois. Messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs. Le Sénat se prononce ce soir sur une proposition de résolution sur l'avenir de l'Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes communément dénommée Frontex. Je voudrais en 1er lieu. Celui du travail de la commission des lois des deux rapporteurs, la personne du président. Et du sénateur Raphaël nous permet de débat de ce soir, du rôle de Frontex agence déterminante pour la maîtrise de nos frontières. Objectif qui passe indiscutablement par une action coordonnée à l'échelle européenne. Certains d'entre vous l'ont déjà rappelé en 2022 la pression migratoire a rejoint un niveau proche d'avant crise sanitaire. Des franchissements irréguliers. Détectés par Frontex aux frontières extérieures ont progressé de 64%. Par rapport à 2021, même s'il reste en deçà de ceux enregistrés pendant la crise migratoire de 2016. Les flux migratoires progresse ainsi dans toute l'Europe. Avec une pression particulière mais il Karen est central dans les Balkans occidentaux. Ce qui fait peser une pression particulière sur l'Autriche, la Hongrie et la Croatie. La demande d'asile a progressé de 61% en Europe. Et de 31% en France, qui reste le second pays d'accueil après l'Allemagne. Tout en étant le premier États à réaliser des transferts. Dublin vers d'autres pays européens. La France reste la cible. Le mouvement secondaire qui traduit la nécessité. De faire évoluer le système européen de l'asile. Mesdames, messieurs les sénateurs. La détermination du gouvernement est totale. Pour apporter des réponses efficaces à cette situation migratoire. Au niveau national. Elle passe par le projet de loi pour contrôler l'immigration. Et améliorer l'intégration qui a été présenté en conseil des ministres. Ce mercredi 1er février par monsieur le ministre de l'intérieur des Outre-Mer et le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Ce projet de loi portera des dispositions inédites. Pour éloigner les étrangers représentaient une menace pour l'ordre public. Pour garantir l'intégration par la langue par le travail par le principe du respect de la République et pour simplifier, très largement. Le contentieux des étrangers Le contentieux des étrangers et une réorganisation de la ville. Le Sénat, Monsieur le Président, aura l'occasion d'examiner ce texte dès le mois de mars. Pour donner des outils juridiques nouveaux à nos dispositifs migratoire. Ces instruments viendront à l'appui des moyens importants, que le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer consacre à la politique migratoire. Il m'importe de rappeler que la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Prévoit notamment la construction de 3000 places de. À l'horizon 2027 pour renforcer notre efficacité. Dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle prévoit également une hausse de 24%. Du budget consacré à l'intégration au cours des 5 prochaines années, en particulier pour l'intégration des réfugiés et pour la maîtrise du français par les étrangers primo-arrivants. Mesdames, messieurs les sénateurs. La ne trafic cité suppose une coordination. Et des politiques communes à l'échelon européen. Il est indispensable de travailler avec nos voisins et une gestion coordonnée c'est-à-dire ordonné des migrations. Comme cela a été reconnu par tous à l'occasion du sommet de La Valette en 2015 et par le Pacte mondial sur les migrations Hadopi manque à Marrakech en 2018. Sous l'égide des Nations-Unies. À la suite du débarquement de l'Océan Viking à Toulon le 11 novembre dernier. La France a demandé et obtenu la tenue d'un conseil extraordinaire des ministre de l'Intérieur qui a permis l'adoption d'un plan d'action européen sur la Méditerranée centrale. Ce plan d'action prévoit notamment une approche mieux coordonnée des sauvetages en mer. Notamment en ce qui concerne l'action des ONG et une coopération renforcée avec les États tiers, sur la prévention des départs irréguliers. La présidence française du Conseil de l'Union européenne a permis par ailleurs de débloquer les négociations sur le pacte sur la migration et l'asile présenté par la Commission européenne en septembre 2020. Grâce à une approche graduelle. La France a réussi à faire progresser les négociations. Dans le cadre d'un juste équilibre fondé sur la responsabilité, la solidarité. Cet accord a été obtenu au Conseil Justice-Affaires intérieures de Luxembourg le 10 juin dernier. Dans le cas des négociations en cours. La France soutient mais Kazim de solidarité contraignant et prévisible pour soulager les pays de la première entrée. Et par des procédures aux frontières extérieures pour lutter contre les mouvements secondaires dans ce cadre. Et c'est dans ce cadre que la France soutient la montée en puissance de l'agence Frontex. Qui est un instrument essentiel. De la protection des frontières européennes et contrôle des flux migratoires. Vous l'avez souligné l'agence Frontex a connu successivement 2 réformes majeures en 2016 et en 2019. Qui ont considérablement élargi le Champ de ses compétences. Règlement de 2019 a permis à Frontex, de passer d'un rôle réactif a un rôle proactif. De prévoir des déploiements à long terme, là où jusqu'alors l'agence ne pouvait que réagir aux situations d'urgence. Frontex est ainsi, il faut le noter, devenue la plus importante agence de l'Union européenne. Dotée d'un budget de 5 6 milliards d'euros pour la période 21 27 et une force prévue à 10.000 agents opérationnels qui pourront être déployés à terme aux frontières extérieures. Et là gît sur plusieurs terrains d'opération Méditerranée. Italie, Grèce, dans l'est de l'Europe à la frontière avec la Biélorussie, mais également dans la Manche. Depuis décembre 21 la Frontex déploie ainsi un avion dédié pour renforcer la capacité de détection. Des tentatives de traversées de migrants par les Small boat sa destination de la Grande-Bretagne. Mesdames, messieurs les sénateurs. La proposition de résolution que vous examinez aujourd'hui. À vocation à conforter le mandat de Frontex à la suite du renouvellement de la gouvernance de l'agence. Le gouvernement partage totalement l'esprit et les grandes orientations de cette résolution. À savoir, elle soutient le renforcement de la veille opérationnel de Frontex dans la surveillance des côtes français et belges de la Manche et de la mer du Nord. Elle encouragent le renforcement du pilotage politique de Frontex. Position porté par la France pendant notre présidence du Conseil de l'Union européenne. Ce pilotage passera notamment par une discussion annuelle du conseil Schengen sur les grandes orientations de l'agence elle soutient le renforcement du rôle de l'agence en matière de retour concrétisé notamment par l'organisation de vols conjoints mutualisant les moyens d'éloignement et d'escorte par les États. Elle propose enfin de laisser le temps à l'agence d'assumer pleinement son mandat actuel sans engager une révision de son règlement position partagée par le gouvernement français. Mesdames, messieurs les sénateurs, l'un des points de cette discussion portera vraisemblablement sur le respect des droits fondamentaux par Frontex dans l'exécution de ses missions. Il me semble. Utile de rappeler ici que Frontex est tenu par son règlement fondateur d'assurer la gestion efficace des frontières. Alors le plein respect des droits fondamentaux. Cet impératif est déjà clairement partie du mandat du nouveau directeur du exécutive exécutif de l'Agence. Dont l'arrivée était accompagné par la nomination de 45 contrôleur des droits fondamentaux et d'un adjoint l'officier aux droits fondamentaux de l'agence. Les allégations de refoulement des migrants en Méditerranée reproché à Frontex ont été traités par plusieurs instances de contrôle. Elles ont conclu que Frontex n'avait pas participé au refoulement. Mais qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'elle n'avait pas eu connaissance de ses agissements. Les recommandations du conseil d'administration de l'Agence du parlement européen de la médiatrice de l'Union européenne ont donné lieu à la mise à la mise en place de plusieurs mécanismes de garantie des droits fondamentaux pour permettre un traitement efficace des signalements des plaintes et des sites et des incidents graves. La France assurera de ce suivi. Dans le cas du conseil d'administration de l'Agence où siègent États. Notre priorité est désormais celle que vous avez soutenu d'accompagner la montée en puissance du corps permanents de Frontex qui doit compter 10.000 hommes en 2027 et auquel la France doit prendre toute sa part. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez compris la question que vous soulevez aujourd'hui au coeur. Des préoccupations migratoire du gouvernement comme elle est au coeur de. Tous nos concitoyens. La question de la maîtrise des flux migratoires et décisive pour la France et pour l'Union européenne. Nous continuerons à agir en ce sens avec des moyens à la hauteur des attentes des Français. Je vous remercie. la. Présidente Nathalie Delattre nous a fait savoir qu'elle était un peu retardé donc elle prendra place dans la suite de la discussion générale. C'est le président, Monsieur le Ministre, messieurs les présidents de des commissions des lois et des affaires européennes sur les rapporteurs. Mes chers collègues. 330.000 c'est le nombre de franchissement irrégulier recensés. En 2022 par Frontex. Aujourd'hui c'est une véritable pression migratoire que subit l'Europe. Et avec elle le risque. D'un bouleversement. Démographique, voire culturel. Ainsi. Au moment où le nouveau directeur exécutif de Frontex. S'installe progressivement dans ses fonctions. Il semble impératif que. En 1er lieu l'agence revienne à son mandat originel. À savoir la surveillance et la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est ce que défend trotte cette proposition de de résolution et nous ne pouvons que. Nous en réjouir. Depuis sa création, Frontex a vu ses missions, ses prérogatives s'accroître considérablement on incluant, par exemple la lutte contre l'immigration illégale. Le trafic de drogue et la criminalité organisée. Cet élargissement des des prérogatives. De l'agence s'est accompagnée. D'une recrudescence d'une recrudescence ces dernières années. Des critiques et des controverses, notamment d'ONG humanitaires. Comme de véritables propagande organe de propagande, opposé à l'idée même de frontières ce qui a considérablement fragilisé l'action de Frontex. Certains l'accusant de ne pas agir suffisamment pour protéger le droit, les droits des migrants. D'autres considérant que Frontex et responsable de la répression excessive des migrants à la frontière. Frontière n'est pas une agence humanitaire et prenons garde à ce qui voudraient transformer cette agence. En un SOS Méditerranée, version 2.0. Car dès lors des milliers de migrants. Arriveront sur des côtes européennes à la merci de passeurs associé au Crime organisé spécialisé dans l'esclavage moderne à travers la traite humaine de malheureux. Les conséquences pourraient être désastreuses. D'un point de vue humain au vu. Des rallyes des réalités démographiques du continent africain. Monsieur le Ministre, face à ces accusations à ces tentatives de déstabilisation. La France se doit de soutenir Frontex dans son mandat et continuer de donner à l'Agence les moyens de sa mission. Frontex. Nous l'avons dit, n'est pas une agence bisounours. Elle est là pour garantir la sécurité et l'étanchéité de nos frontières européennes. Pour se fier il faut éloigner les ONG. Les agences humanitaires de contexte et remettre les pays souverain au centre. Des choix de l'agence. Mais il faut veiller bien évidemment à ce que Frontex agissent de manière responsable et respectueuse des droits de l'homme. Et prenons garde car à laisser l'angélisme irresponsable dicter notre politique migratoire commune, nous prêtons le flan au populisme et à l'extrémisme qui n'attend qu'un écart de notre part pour mettre à mort le projet européen, ce qui constituerait un recul sans précédent pour l'enfant. La France et l'ensemble des États membres. Alors, ne cédons pas aux injonctions de la bien pensance qui nous adresse toujours le même message, celui qui se veut Angélique mais qui est en réalité inconscient. Liberté pour les migrants et honte aux frontières. Mais la France est généreuse. Et elle n'est pas J. mosaïque de territoire sans limite, c'est une nation en droit de choisir qui peut la rejoindre en droit aussi d'exiger des étrangers qu'ils se plient à ses règles, à ses coutumes et à sa culture, c'est pour cela que la France ne peut s'exonérer de sa propre politique migratoire la double souveraineté nationale et européenne et complémentaire ne cachons pas la poussière migratoire sous le tapis européens en fermant les yeux sur ce sujet, Monsieur le Ministre le en même temps. Conduit à l'impuissance et donc à l'échec ne détournons pas le regard engageons-nous résolument sur ces 2 niveaux de souveraineté pour apporter une réponse totale. Une réponse à 360 degrés pour contrôler nos frontières. C'est notre ambition. Avec le projet de loi immigration qui arrive prochainement au Sénat, nous aurons l'occasion de débattre et de bâtir une réelle politique de maîtrise de notre souveraineté migratoire française et européenne car c'est là le coeur de toute nation la maîtrise du cours de son destin merci. Merci cher collègue. La parole est maintenant monsieur Franck Menonville pour les indépendants et pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Madame et messieurs les présidents. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Les confinements des dernières années ont mis un coup d'arrêt brutal à la circulation des personnes. La pandémie est désormais sous contrôle et les déplacements de population ont repris. Qu'ils soient légaux ou non ils sont à présent en pleine expansion. C'est ainsi que l'Union européenne dénombre pour l'année 2022. Environ 330.000 franchissement irrégulier de notre frontière commune. La prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan le chaos libyen ou encore celui de Syrie. Constitue et continue d'alimenter ces mouvements de population. En 2015 déjà, l'Europe avait connu une crise migratoire majeure. L'Union avait déjà délégué le contrôle de ses frontières à la Turquie d'Erdogan qui s'étaient empressés de l'utiliser comme un formidable moyen de pression. Avec nos partenaires européens nous prenions à Lyon alors conscience. Que si la libre circulation en Europe est une chance. Elle constitue également une vulnérabilité majeure si les frontières extérieures si la frontière extérieure En 2014 le budget de Frontex agence en charge de contribuer à ce contrôle s'élevait à 93. Millions d'euros. Moins de 10 ans plus tard, ce budget a été multiplié par 9. Prenant conscience de la valeur de la mission confiée à cette agence. Les États membres lui ont confié donc les moyens les plus importants qu'une agence européenne n'ait jamais eu. D'ici 4 ans. Elle devrait ainsi voir ses effectifs opérationnels atteindre 10.000 agents. Les temps futurs s'annonce difficile, les cris géopolitiques se multiplient. Les manoeuvres biélorusse du de de novembre 2021 nous rappelle que les flux migratoires peuvent être employé comme des armes de déstabilisation. Il nous faut donc augmenter les moyens consacrés à la surveillance de nos frontières. Nous allons en avoir besoin. L'agence Frontex rencontrent des difficultés dans l'accomplissement de sa mission. Cela tient principalement au fait qu'elle doit à la fois bien évidemment protéger les frontières européennes. sans laisser porter atteinte aux droits fondamentaux des migrants et c'est essentiel. L'Union européenne puissance normative ne peut pas admettre que le droit soit bafoué. La résolution que nous examinons aujourd'hui nous semble tout à fait équilibrée et nécessaire. Nous partageons le souhait de saluer le travail de Frontex et la volonté de lui témoigner notre confiance. Nous appelons donc au renforcement de ses moyens. la présente résolution est examinée en séance publique, car le groupe geste et socialistes ont tenu à exprimer leur préoccupation quant au respect des droits font demain autour des des migrants. Ces préoccupations sont légitimes mais nous pensons qu'il faut pas perdre de vue la raison d'être de Frontex. La surveillance des frontières européennes. Si la Grèce a procédé à des à des refoulements illégaux si la Pologne n'a pas souhaité faire appel à Frontex afin d'avoir les coudées franches. Si la Hongrie a construit un mur de barbelés. Si le Royaume-Uni et le Danemark ont envisagé de renvoyer leurs migrants vers le Rwanda. Si l'extrême droite est au pouvoir en Italie et qu'elle pourrait être demain dans d'autres pays européens, c'est bien le signe que quelque chose ne va pas dans notre pays, nous devons disposer d'un d'une véritable politique migratoire qui s'appuie sur le socle des valeurs républicaines que sont notamment la maîtrise de la langue, vous l'avez évoqué, monsieur le Ministre, la laïcité ou encore l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une attente légitime de nos concitoyens. les politiques migratoire plus stricte menés par le Danemark doivent nous inspirer en effet la situation migratoire européenne n'est plus acceptée par nos concitoyens, et il est urgent d'agir. Il sera sans doute indispensable à terme de revoir nos procédures pour faire respecter à la fois notre droit, tant en matière de droits fondamentaux qu'en matière d'entrée sur le territoire européen. Pour l'heure, nous pensons qu'il faut laisser à Frontex. Le temps de monter en puissance et d'intégrer les nouvelles composantes qui lui ont été adjointe un contrôle politique nous paraît essentiel car c'est aux politiques de prendre les décisions et d'en assumer les conséquences. Par conséquent le le groupe les impôts dépendant votera en faveur de cette résolution. Merci. Merci. Rien. Maintenant, la parole est à monsieur Jacques Fernique. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires et pour cinq minutes également. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Au cours des 6 mois de présidence française du Conseil. Le gouvernement avait comme objectif de rendre l'Europe plus humaine. Mais entre les slogans et les actes on constate. Un peu toujours le même fossé certes l'Union ces États. Ses citoyens ont fait preuve d'une générosité d'une solidarité sans faille pour accueillir les ukrainiennes et ukrainiens. Mais dans le même temps la la France plaidait au Conseil pour le renforcement du contrôle des personnes aux frontières de l'Union à travers le règlement sur le filtrage et une surveillance accrue par le renforcement de la base de données biométriques Eurodac. La solidarité contrairement au dispositif de répression n'a fait l'objet que d'une déclaration non contraignant. Mes collègues eurodéputés du groupe écologiste ont observé au niveau européen une continuité de la ligne disons-le brutale suivie tout au long du précédent quinquennat. Celle de la loi Asile et immigration. 2018. La guerre en Ukraine, quant à elle a démontré qu'il est possible d'accueillir des exilés avec dignité. C'est la première fois que la directive protection temporaire datant de 2001 était activé. Les autres irakiens, afghans syriens on les affuble du terme de migrants plutôt que celui de réfugié leur parcours migratoire et souvent criminaliser qui sont solidaires aussi ainsi Mimmo Lucano en est un exemple frappant alors qu'il a fait le choix d'accueillir dignement des exilés dans le petit village de Calabre, dont il était maire, il risque aujourd'hui jusqu'à 13 ans de prison. Je crois qu'il faut s'interroger avec clairvoyance sur les causes et les mécanismes des flux migratoires. Regardons la situation en face. 87% des migrations dans le monde se font dans le pays voisin de celui qu'on a fui. Seule une petite partie de ces personnes demandent à être accueillis dans l'Union européenne mais depuis des années, notre Union européenne à traiter les questions migratoires principalement par une surenchère sécuritaire. C'est pas un succès, c'est plutôt une défaite est une défaite morale. Je crois qu'il est temps de proposer un pacte sur la migration et l'asile à la hauteur de l'exigence humanitaire. Il y a des femmes, il y a des enfants il y a des hommes qui meurent à nos frontières chaque jour personne ne peut dire qu'il ne sait pas. Frontex. Mais de fait. En péril la bonne conduite des opérations de sauvetage et de secours en mer par les navires affrétés par des ONG, des situations humanitaires intenable en sont le résultat, on a parlé d'Océan Viking, en 2022 et même lorsqu'ils ont débarqué sur le sol européen. Les exilés ne voient pas leurs droits les plus fondamentaux correctement reconnus. Comme le demande mes collègues écologistes au Parlement européen, les 900 millions d'argent public finançant Frontex. On a parlé pour la période 2021 2027, de 5 6 milliards. Une partie pourrait servir à financer une vraie politique de contrôle et d'accueil à grand budget grande responsabilité Frontex doit agir avec plus de transparence et cesser d'ignorer les demandes légitimes formulées par les eurodéputés. Ce qui se passe aux frontières de l'Union et hélas bien trop souvent la négation de la dignité humaine, et cela se passe, c'est passé avec la passivité, voire le concours de Frontex et je ne décèle pas dans cette résolution de, de volonté d'y mettre un terme. J'y vois surtout un vocabulaire d'un Champ lexical plutôt militaire sécurité menace anticipation des risques criminalité. On y parle certes de potentielles irrégularités alors que c'est quand même d'importants manquements dysfonctionnements qui ont été mises à jour et dénoncé. Par l'Office européen de lutte antifraude, le Parlement européen des ONG, les journalistes dans cette proposition de résolution la garantie du respect des droits humains apparaît à la fin d'une phrase ou est souvent systématiquement minoré d'un mais. Ces 48.647 personnes qui sont mortes aux frontières de l'UE depuis 93. Ce bilan n'est mentionné nulle part dans la résolution. Combien. Ce soir l'ont évoqué, depuis le début de ce mandat. Cette résolution, elle estime qu'il est nécessaire de laisser à Frontex. Le temps de mettre en oeuvre l'intégralité de son mandat actuel or permettent à Frontex de continuer avec les mêmes règles. C'est, je le crains conforter des violations du droit européen et international et je pense que dans ce contexte, la France devrait plaider au Conseil pour une refonte structurelle et complète de l'agence et non pas simplement pour repousser la date butoir. Via cette résolution nous aurions pu aussi nous Sénat envoyer un signal politique fort, comme l'a fait. Le Parlement européen en refusant de voter la décharge budgétaire des euro-députés de tous bords ont exigé une rupture dans la culture interne et la pratique de l'agence nous croyons profondément la capacité collective de faire des choix de solidarité. C'est le sens de nos amendements qu'ils s'ils étaient Merci, cher collègue, la parole maintenant Madame, Patricia Schillinger pour le groupe RDPI. Et pour six minutes.

Schengen, la liberté de circulation est au coeur du projet de l'Union européenne et le rôle de l'agence Frontex, créée en 2004 et de veiller à ce que nos frontières extérieures remplissent pleinement leurs fonctions. La France est convaincu de la pertinence d'un engagement de Frontex lorsque États est confronté à des difficultés à ses frontières extérieures car celles-ci sont les frontières de l'UE et justifie une réponse européenne depuis 2015, la crise migratoire et de la ville à laquelle a été confrontée l'Union européenne a provoqué une importante réforme de l'agence Frontex conduisant à l'augmentation de ses missions et de ses moyens. Une première extension de son mandat la conforter en tant que bras opérationnel de l'Union européenne. Acteur de 1er plan de la politique migratoire européenne mais depuis 2015, les flux n'ont cessé d'augmenter et les derniers chiffres en témoignent, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté de en 2022 de 64% par rapport à l'année précédente, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016, soit 330.000 entrées irrégulières enregistré en 2022 dont 45% sur la route des Balkans. Face à ces flux. L'agence a dû procéder non pas sans difficulté à des profondes transformations dans des délais restreints et construire notamment des capacités opérationnelles autonomes comme ici même au Sénat, l'ancienne directrice par intérim de l'agence en effet dans un contexte international crispé marquée par la pandémie de Covid. Covid-19, l'instrumentalisation des flux migratoires par la Biélorussie, en novembre 2000, maintien ou le déclenchement du conflit en Ukraine en février 2022, Frontex a été soumis à rude épreuve et a traversé une véritable crise de croissance depuis ses capacités opérationnelles ont été décuplées avec une montée en puissance rapide et massive des moyens matériels, notamment avec un budget de 845 millions d'euros en 2023. Dans le même temps et comme l'ont souligné nos présidents François Noël Buffet et Jean-François Rapin, que je remercie pour la qualité de leurs travaux. L'agence a fait l'objet de nombreuses accusations concernant aussi bien le respect des droits de l'homme que le. Que les refoulements la mauvaise gestion interne ou encore les conflits personnels au sein de l'agence, une crise de confiance qui a ébranlé le sérieux de l'Agence auprès de l'institution européenne et des États au au regard de ces crises de croissance et de confiance. La Commission européenne envisage de réviser le règlement européen et qui défini le mandat de Frontex. Ce que nous souhaitons, ce que nous ne souhaitons pas dans l'immédiat. À l'instar de la proposition de résolution examiné aujourd'hui dans la mesure où l'agence n'a pas encore pu absorber les derniers et élargissement de son mandat. Toute nouvelle révision serait prématurée. Nous soutenons également le triple objectif soutenu par nos collègues dans cette proposition de résolution objectif à la fois politiques, diplomatiques et juridiques qui commande un renforcement du pilotage politique de la redevance des représentants qualifiés par l'État membre au sein du conseil d'administration, une évaluation rigoureuse de l'officier aux droits fondamentaux. Ce soutien ne doit pas nous mettre et il exige une clarification forte de l'agence quant au respect des droits fondamentaux dans le cadre de ses missions ainsi que soit associé les parlements nationaux dans le contrôle de l'agence. À ce titre, la mise en place d'un groupe de contrôle parlementaire conjoint sur le modèle de celui établi pour contrôler les activités d'Europol nous semble être une piste sérieuse a envisagé nous émettons enfin une observation sur le regret exprimé par le PPR concernant le choix du gouvernement français à s'abstenir de désigner un candidat au poste de directeur exécutif, nous tenons à souligner que l'influence française est encore présente et porte ses fruits. La France a soutenu la nomination à la tête de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information EI et la Française Agnès Diallo après l'intérim de Luca Taghlit Harry, chers collègues, cette observation faite nous soutenons pleinement cette proposition de résolution qui a pour ambition de faire de Frontex une agence tourné vers l'avenir. Doté d'un vrai cap politique d'une gouvernance plus saines d'objectifs clairs et surtout qui s'inscrit dans le respect des droits fondamentaux. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent. Jean-Yves Leconte. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, et pour 9 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le président, mes chers collègues. Lorsque, en 1995. L'espace Schengen a été mis en oeuvre. Posant le principe dans cet espace de la liberté de. Circulation sans contrôle aux frontières intérieures. Nous avions à leur poser le principe que chaque État. Membre de cet espace était responsable de sa partie de frontière extérieure de l'espace Schengen. Bien entendu, des échanges, des échanges d'informations ont été mis en place une part à un partage de la politique de visas de court séjour. Une des politiques d'asile concertée conjugués ont été mis en oeuvre mais nous nous sommes arrêtés là et puis il y a eu l'élargissement de 2004 la mise en place de Frontex principalement pour surveiller les nouvelles frontières de l'Union européenne. Et puis 2015 Le terrorisme lié à l'avènement de Daech aux portes de l'Europe. Et que nous avons vécue dans notre Chair en France et à Paris. La guerre au Proche-Orient la guerre en Syrie qui a jeté des millions de personnes sur les routes de l'exil à l'envers l'Europe. Notre construction européenne conçue dans un océan calme n'était plus adéquate. C'est la raison pour laquelle a été mis en place à partir de 2016 un certain nombre de nouveaux projets. Le système entré Schengen entrée sortie biométrique qui va être progressivement mis en place le projet Ethias et aussi le nouveau mandat de Frontex en 2002 1016 mandat Frontex qui a conduit à constater que que 1er budget de Frontex supérieur à 100 millions d'euros en 2015. En 2023, le budget 845 millions d'euros. Entre 2018 et 2027, il va y avoir plus qu'un doublement du contingent permanent chargé pour Frontex. Voilà ce qui a été fait, ce qui a été mis en oeuvre pour préserver la liberté de circulation dans l'espace Schengen, la sécurité de l'espace Schengen et. Cette ces évolutions. Nous constatons qu'effectivement. Ça a provoqué auprès de Frontex finalement de de de de situations, d'abord ça a été déjà dit une crise de croissance gérer en quelques années une multiplication par plus que 8 des Budgets une multiplication par plus que trois du nombre de personnes qui étaient. De du du contingent Frontex et de nouvelles responsabilités et puis je dirais une crise plus plus systémique et qui n'est pas résolu. Le fait que Frontex contrairement à son nom n'est pas le garde-frontières de l'Union européenne Frontex est une agence d'une certaine manière un prestataire de service au service d'état qui maintienne l'ensemble de l'eau sous leur souveraineté à chaque partie de frontières extérieures de l'espace Schengen, une espèce de l'Union européenne et c'est finalement la difficulté de de 2 exemples. Le 1er ce qui s'est passé entre la Pologne et la Biélorussie. L'année dernière. À l'été à l'Automne 2021. Une situation tout à fait nouvelle et inattendue. D'arrivées de migrants en provenance de Biélorussie vers les frontières de la Pologne et de de de la Lituanie, la Pologne n'a pas souhaité faire appel à Frontex. La Pologne a gérer seul une situation. Dans une situation profondément. Choquante par rapport au respect des des droits fondamentaux. Aucune transparence aucune capacité pour les journalistes ou les parlementaires du pays de voir ce qui se passait dans la zone frontalière, ce sont les témoignages des habitants de cette zone qui permettent de savoir aujourd'hui comment la situation a été réglé par la Pologne mais la Pologne n'a pas fait appel à Frontex. Parce que Frontex. avait et a des exigences en matière de droits fondamentaux. Et quand tu. 2ème exemple la Grèce. En 2021, un certain nombre de médias, un certain nombre d'ONG ont fait part de push Back. Sur terre et sur mer. De migrants arrivant en Grèce et qui ont été refoulés de manière absolument scandaleuse. Frontex. Ah vu ces situations. Mais Frontex agit toujours sous la responsabilité de l'État membre. La difficulté c'est que si en 2016, nous avons choisi de donner un nouveau mandat à Frontex. C'est justement en particulier pour faire face à la situation pour accompagner la situation aux frontières sud de l'Union européenne et en Grèce. Alors bien entendu, si. Nous disons. Nous dénonçons ce qui s'est passé aux frontières entre la Grèce et la Turquie, ça remet aussi en cause. La capacité de Frontex de continuer à agir en Grèce et c'est toute la difficulté Frontex aujourd'hui ne peut pas remettre en cause. Un certain nombre d'États qui sont finalement. Fondamentaux. Et qui doivent avoir besoin de Frontex et c'est bien la situation que nous avons avec la Grèce. Comment voulez-vous remettre en cause si si si la Grèce Mendy. Écoutez, on ne veut plus de Frontex. Comment vont être pour surveiller les frontières.

Hé bien il faut être intransigeant sur le respect des droits fondamentaux par Frontex et il faut faire en sorte que, au sein de Frontex et c'est ce qui. Ce que ce que la crise finalement de 2021 2022 de Frontex a essayé de mettre en oeuvre une plus grande indépendance de personnes chargées de respecter les droits fondamentaux à l'intérieur de l'agence de manière à ce que finalement ce soit pas le le le le la responsabilité exclusive du directeur de Frontex de s'assurer que Frontex. Soit. Irréprochable en matière de droits fantôme et les droits fondamentaux. C'est pas une option, c'est une condition de l'efficacité, c'est une condition de la crédibilité parce que Frontex doit aussi intervenir hors de l'Union européenne Frontex peut aussi intervenir. dans des pays européens comme par exemple la Macédoine ou la Moldavie et Frontex peut peut être dans certains sont de cas être amené à accompagner un certain nombre de pays, au sud de la Méditerranée pour surveiller les frontières. Mais pour cela il faut que Frontex soit Or ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui et la raison de la condition de l'efficacité de Frontex. C'est bien d'avoir une surveillance interne en matière de respect des droits fondamentaux qui est d'un autre niveau que ce qui existait jusqu'à présent et que ce qui est posée par la proposition de résolution. Alors c'est la raison pour laquelle, même si nous partageons. La volonté d'un plus fort pilotage politique du Conseil de de de Frontex par son conseil d'administration avec un conseil d'administration, plus politique, même si nous partageons la volonté et le constat de dire que le mandat de Frontex doit être. Pleinement développée et pleinement mis en oeuvre avant de penser à un nouveau mandat. Même si nous partageons la volonté d'avoir un contrôle des Parlements nationaux plus fort. Nous ne pouvons pas aller et accompagner la proposition de résolution. Sans que nos amendements soient adoptés car nous considérons que sur. La question des droits fondamentaux. La proposition de résolution ne va pas assez loin. Il est absolument essentiel que la protection et l'observation du respect des droits fondamentaux par Frontex et dans les opérations ou Frontex participent soit irréprochable et surveiller de manière indépendante. C'est la raison pour laquelle nous poserons trois amendements qui, si elles étaient adoptées nous permettrait d'accompagner. Cette proposition de résolution dont vous avez compris que nous partageons l'essentiel parce que Frontex est un élément essentiel pour garantir la liberté de circulation dans l'espace Schengen pour garantir notre politique. De surveillance des frontières, mais nous ne pouvons pas accepter que Frontex ne soient pas surveillées de manière irréprochable et ne soient pas irréprochable en matière de droits fondamentaux, que ce soit, directement ou dans les opérations conjointes. Avec un certes avec les États, parce que si Frontex intervient Frontex doit intervenir dans des opérations qui sont irréprochables. De cette manière-là et ce n'est qu'en garantissant l'indépendance totale de ce qui dans l'agence hausse chargé de cette surveillance que nous pourrons garantir que Frontex soit à la fois irréprochable et donc efficaces sur le long terme, c'est la raison pour laquelle nous proposerons des amendements pour être en mesure d'adopter cette proposition de résolution sinon malheureusement nous ne pourrons pas vous accompagner, même si sur les autres sont. Objectif, nous sommes d'accord. Merci, cher collègue, la parole est à présent au président Pierre Laurent pour le groupe CRCE. Et pour cinq minutes. Selon le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons nous prononcer ce soir sur une proposition de résolution européenne vivant les missions de l'agence Frontex, dont l'action a été serveur sévèrement mis en cause la résolution vise à lancer un message de soutien à l'agence après ces mises en cause. Elle évoque certes les graves 10 accusations de manquement au respect des droits fondamentaux. Comment pourrait-il en être autrement après les constats dressés par le Parlement européen et le rapport de l'Olaf. Mais force est de constater qu'elle minimise grandement les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer. Les recommandations qu'elle énonce en matière de relance et de gouvernance de l'Agence semblent toutes encadrées par l'obsession alarmiste de la situation aux frontières extérieures de l'Europe. En parlant de crise de croissance comme facteur explicatif la résolution évacue tout lien entre les dérives constatées et la conception même des missions confiées à Frontex. Or c'est bien là qu'il conviendrait de Touré interrogé car la dérive vers la mi-la militarisation de fête des frontières de l'espace Schengen a partie liée à une politique de plus en plus. Restrictive à l'égard de l'accueil et à l'égard du respect du droit d'asile, dans lesquels s'enracine les dérives constatées portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes migrantes. Désormais balafré de 19 conclure clôture frontalière sur plus de 2048 Schengen prend toujours plus des allures d'une forteresse qu'il s'agirait de défendre par tous les moyens. Le texte évoque par exemple l'efficacité du partenariat entre la Grèce et Frontex. Or, faut-il rappeler le rapport de l'Olaf pointant précisément la complicité de l'agence dont l'abandon par les autorités grecques de groupe de migrants sur de petits îlots inhabitable. Par la militarisation de ces. De ces agents Frontex est le symbole du prolongement de la réticence des États européens à appliquer le droit des îles et une politique d'accueil digne. Faute d'une politique européenne à la à la hauteur de nos devoirs d'accueil et de solidarité humaine. C'est en vérité une véritable crise humanitaire qui sévit chaque jour aux frontières de l'Europe. Des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants se noient toujours en Méditerranée. Ou meurt d'hypothermie dans l'est de l'Europe, des femmes victimes de violences poussé sur les routes de la migration par des réseaux de traite sont refoulés sans ménagement. Des mineurs sont aussi refoulé en bafouant le droit international. Malgré cette militarisation progressive de Frontex, la multiplication de son budget par 17 depuis sa création 2004 aucun effet dissuasif n'est par ailleurs constaté. de, de sol, des politiques de migration concertée, organisée autour de voie légale et sécurisée permettant des parcours respectueux des droits fondamentaux des personnes seraient à même de changer la situation, nous percevons-nous persévérant dans l'inhumanité ériger des murs toujours plus haut externaliser la gestion des frontières extérieures sans jamais ni tarir les causes des migrations subi ou forcer ni en finir avec les refoulements expéditifs les politiques répressives en vérité n'arrête pas les migrations elle légalise l'arbitraire les clôtures, les barbelés, les barrages de toute nature. Un accueil digne réclamée à cor et à cri par les gouvernements les plus à droite ou à l'extrême droite en Europe ne font qu'en réalité que favoriser l'insécurité les contournements l'émigration irrégulière frontière ex- devient le bras armé de ces politiques quand elle devrait assister au contraire les États dans une gestion humaine digne et sur des frontières à l'échelle européenne. La démission de l'ancien directeur exécutif de Frontex n'a été en vérité qu'un symptôme d'un mal profond celui d'une activité aux frontières gangrénée par la dissimulation de violations commis par des États membres de l'UE en matière de droits des migrants. Il apparaît de plus en plus évident que Frontex manque cruellement de mécanisme de responsabilités, tant au sein de l'agence qu'à l'extérieur. Une préoccupation que la résolution semble réprimer comme si un contrôle effectif et indépendant en matière de respect des droits fondamentaux serait synonyme de frein dans la mission de Frontex. Dans ces conditions, laisser Frontex aller au bout de son mandat s'en remettre à plat par une évaluation approfondie ses missions et les politiques qui les sous-tendent nous paraît au minimum bien insuffisants au regard des graves manquements constatés comme des objectifs non atteints en matière de responsabilisation des États membres, dans le respect des droits fondamentaux et du droit européen. Cela ne nous semble pas raisonnable. C'est entre autres pour cette raison pour cette conclusion de la résolution qui ne court qu'elle qui nous conduira pardon a voté contre cette résolution. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Jean Michel Arnaud pour le groupe Union centriste. Et il dispose de 8 minutes. Monsieur le président. Monsieur le ministre, messieurs les présidents des commissions. Monsieur le rapporteur. Chers Arnaud. Mes chers collègues. Cette proposition de résolution nous permet de mettre en lumière le sujet brûlant des migrations vers notre Europe toujours Mercier à cet effet. Les collègues socialistes écologistes de nous donner l'occasion d'en débattre publiquement ici en séance ce soir. Les défis de l'Europe face au flux migratoires 50 bel et bien à travers les récentes mutations non sans difficulté de l'Agence européenne des gardes-frontières et gardes-côtes 10 Frontex. Comme cela a été rappelé cette agence sans doute la plus connue de nos concitoyens. Une triple mission, assurer un rôle de veille permanente aux frontières extérieures de l'Union. Être en appui des États, dans la lutte contre la criminalité. Transfrontalière et aider les pays tiers et ont passé un accord avec l'Union européenne à juguler les flux migratoires irréguliers vers l'Europe. Jamais une agence supranational ne s'est vu conférer de telle prérogative de puissance publique. C'est mission ayant été renforcée en 2016 et 2019. Ce sont également accompagnés d'une allocution. Accrue. Des moyens humains et financiers 5 8 milliards d'euros seront mobilisés dans les années à venir, avec l'objectif d'atteindre 10.000 personnels à l'horizon 2027 qui soit propre à l'institution ou détaché des États membres. Cette volonté de faire de Frontex, l'apanage de la politique migratoire européenne s'est heurtée à de multiples complexité. La croissance fulgurante des moyens dans un temps très court, n'a pas laissé un délai suffisant au bon calibrage de l'organisation, notamment pendant la période de crise sanitaire. Rapport spécial également de la Cour des comptes de l'Union européenne publié en juin 2021 et celui de l'Office européen de lutte antifraude, paru en février 2022 ont mis à mal la légitimité de Frontex. Manque de transparence dans le coût des opérations mais également manquements à des, à ses obligations en matière de respect des droits fondamentaux, comme cela a été rappelé par les collègues. Cumul aux critiques de certains États membres. Ces révélations ont entraîné la démission du directeur de l'époque, Fabrice Leggeri. Enfin ces états de faits ont laissé transparaître des luttes d'influence interne aux institutions européennes. Concernant la politique migratoire entre la protection des droits fondamentaux des migrants. La lutte contre l'immigration irrégulière. Les positions des États membres diverses sur des priorités opérationnel de Frontex. Une clarification de ces missions s'avérait donc nécessaire. L'agence Frontex fait face à une transformation de son organisation, tout en subissant un déficit de légitimité. Alors que ses responsabilités tente à se renforcer. Pour reprendre les termes utilisés par le président de la commission des lois en commission. Ces crises de croissance et de confiance. Appel à proposer un ensemble de recommandations concernant l'avenir de l'agence. Telle est l'objet de la proposition de résolution que nous examinons ce soir j'en profite pour féliciter le rapporteur Jean-François Rapin et Didier Marie pour la qualité de leur travail auxquels j'associe naturellement Arnaud de Belenet pour la commission des lois. Le pilotage politique de Frontex a montré ses faiblesses en effet la récente nomination du nouveau directeur doit s'accompagner d'un conseil d'administration doté de personnel d'une expérience et de niveaux hiérarchiques suffisante. Ainsi la constitution d'un groupe parlementaire conjoint entre les parlements nationaux et le Parlement européen semble indispensable le contrôle parlementaire ne peut être qu'un atout. Il s'agit, tant au niveau du Parlement européen que des parlements nationaux d'assurer une stabilité institutionnelle et une légitimité politique au bénéfice d'organisation en plein développement. Ensuite, le mandat de Frontex se doit d'être également clarifier, telle est l'objet des alinéas 37 et 46 de la proposition de résolution européenne que nous étudions ce soir. La mise en place de certains critères de recrutement pour les contrôleurs aux droits fondamentaux et surtout pour l'officier aux droits fondamentaux est un impératif. Un prérequis en terme d'expérience professionnelle dans le domaine des droits fondamentaux semblent également pertinent. C'est la raison pour laquelle notre groupe soutient vivement cette recommandation visant à soumettre les décisions de l'officier des droits fondamentaux à un avis annuel du médiateur européen. Concernant les opérations conjointes entre l'agence et des États membres. Ces dernières se réalise exclusivement à la demande d'un État et sous l'autorité de ce dernier. Bien que le rôle de l'agence Frontex n'est en aucun cas de surveiller l'action d'un État souverain. Une procédure d'alerte pour violation des droits fondamentaux demeurent en recours, sous réserve que les modalités de de déclenchement de celle-ci soit encadrée. Ça été rappelé également c'est un, un élément majeur pour renforcer la confiance que l'on doit à Frontex mobilisés notamment par des États membres parfois peu scrupuleux en matière d'accompagnement et dignité à l'égard des personnes migrantes. La proposition de résolution européenne appelle aussi au maintien d'une capacité opérationnelle. Si les effectifs s'accroissent la montée en puissance de Frontex doit aller de Pair avec une plus grande train transparence sur l'impact et le coût des opérations et aussi un renforcement des coopérations avec les États membres et des structures communautaires, je profite également de la présence à la tribune ce soir pour appeler une coopération intercommunale plus étroite sur les questions d'émigration secondaire mon département les Hautes-Alpes qui se situe pour ceux qui l'ignoreraient, à la frontière italienne est particulièrement concernée. Entre 2019 et 2020 plus de 11.000 passages illégaux par an ont été répertoriés entre l'Italie et la vallée de Briançon. Ces passages s'effectue principalement via le triste célèbre col de l'échelle, malgré sa beauté cette route extrêmement dangereuse et fermé en hiver. Elle est utilisée également par des passeurs mais aussi par un certains nombres de personnes migrantes et on se pour souci simplement d'avoir un chemin est une destination horizon plus heureux ces désespérés sont parfois aussi victimes de la mort durant les périodes d'hiver. On évoquait tout à l'heure les situations plutôt à l'aise de l'Europe mais également chez nous en France ces situations peuvent se produire la pression migratoire locale et renforcé également par l'inadéquation des moyens alloués à la police aux frontières qui ne permet pas toujours d'assurer correctement leur mission. Pas plus d'ailleurs je le dis au passage que les moyens mis à la disposition des associations humanitaires dans cette ville de Briançon sont à la hauteur de l'accompagnement nécessaire en matière de dignité pour les personnes migrantes prise en charge en urgence. Par cette résolution, je crois pouvoir dire que le Sénat appelle donc nos démocraties européennes à être à la hauteur de leurs idéaux. Nous ne pouvons rester indifférent face à ses enfants à ces femmes à ces hommes qui aspirent à un avenir meilleur en franchissant nos frontières extérieures, mais aussi je viens de leur donner. Démonstration pour la France aux frontières intérieures. Mais nous ne ne vont pas être pour autant naïfs. Le nouveau directeur exécutif de Frontex s'est engagé voici quelques jours à rétablir la confiance dans cette agence européenne de garde-frontières a réorganisé la la façon de fonctionner Frontex et de réduire et de produire pardon des résultats tangibles atteint notamment en termes humanitaires et en respect des droits fondamentaux. Je pense effectivement qu'il est nécessaire que Frontex joue ému dans cette direction afin que l'équilibre soit trouvé entre la nécessité de ne pas être preuve de naïveté à nos frontières face à d'immigration parfois organisée par des réseaux, mais aussi la nécessaire dignité et l'accompagnement en humanité d'un certain nombre de personnes qui ont fait le choix parfois politiques souvent économique et social de venir trouver d'autres espérance vers les frontières européennes, mes chers collègues. Comme vous le d'imaginer. Groupe Union centriste dans ce souci d'équilibre, opère un an qui est le sien votera en faveur de cette proposition de résolution européenne tout encore évidemment cet objectif de d'humanité renforcée en direction des populations les plus fragiles qui arrive en Europe. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame. Esther Benbassa. Au titre des sénateurs n'appartenant à aucun goût. Et elle dispose de 3 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en février 2022, l'ONU a alerté l'Europe contre une normalisation du refoulement illégal des réfugiés à nos frontières. Le rapport de l'ONG Human Rights Watch est accablant à l'égard de l'agence européenne Frontex. La surveillance aérienne exercée par celle-ci permet aux gardes-côtes libyens d'intercepter des bateaux de migrants. Ces derniers sont renvoyés de force en Libye et sont confrontés à la violence, à des abus à l'esclavage et à la torture. Ces faits sont directement imputés à Frontex qui devient alors complice d'actes inhumains. Également un rapport, cette fois-ci de l'Office européen de lutte antifraude dénonce des actes similaires impliquant des agences de Frontex en Albanie et à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Nous ne pouvons fermer les yeux sur ces révélations avec des preuves à l'appui et faire comme si notre soutien à Frontex devait primer sur nos principes fondamentaux. Je ne partage pas vraiment l'avis des rapporteurs pour qui la mission première de Frontex serait de garantir le contrôle efficace des frontières extérieures de l'Europe à des fins de lutte contre l'immigration clandestine. Le respect des droits de l'homme doit dépasser toute considération idéologique et doit être la boussole de nos actions. Les tragédies se succèdent, celle de lampes En 2013, le naufrage de plus de 800 migrants en 2015 celui de 27 migrants dans la Manche l'année dernière et enfin la mort d'une trentaine de migrants depuis le début de l'année en mer Méditerranée. Nous devons prendre toute la mesure de la gravité de l'échec de Frontex dans ses missions. D'après les chiffres de l'Agence européenne 330.000 entrées irrégulières ont été enregistrés en 2022 en Europe. Le système en place est incapable de répondre à la problématique migratoire qui traverse l'Europe en ville en 10%, de ses entrées irrégulières. Sont des femmes et environ 9% des mineurs. Séminal je les ai rencontrés. Au campement de la porte d'Ivry, 400 adolescents livrés à eux-mêmes dans des tentes d'infortune et les exemples sont nombreux. Est-ce vraiment digne de la France. L'Union européenne souhaite remettre la migration au sommet de ses priorités. Il est urgent de réformer Frontex sa mission de contrôle doit être indissociable de sa mission de protection des droits fondamentaux. La Grèce, la Pologne, la Bulgarie, quant à elle réclame le financement européen d'un mur anti-migrants et de barbelés érigée le long de leur frontière l'échéance des élections européennes arrivent à grands pas hélas sans un système d'asile et de migration harmoniser effort je crains qu'une nouvelle poussée des extrêmes surgissent lors des résultats du sceau du suffrage. Je voterai contre ce texte. Merci, Merci, cher collègue, la parole est à maintenant à Madame Catherine Bell Rithy. Pour le groupe des Républicains et elle a 7 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, que resterait-il des frontières de l'Union européenne sans l'agence européenne de garde-frontières et de gardes-côtes appelée Frontex. Aujourd'hui plus que jamais c'est une responsabilité commune que le surveiller d'entretenir les frontières extérieures de l'Union européenne. En 1er lieu Frontex. C'est d'abord indispensable compte tenu de sa raison d'être. La connaissance et la régulation des flux migratoires aux portes de l'Union européenne, il faut le rappeler, car elle doit rester le centre de gravité de nos débats. Chaque événement international de ces dernières années a effectivement conduit à un accroissement de ces flux. Pour n'en citer que 3 exemples issus des années les plus récentes en 2019 2020. Les tensions entre la Turquie et l'Union européenne se sont concrètement traduite par des pressions étrangères sur les autorités locales de Frontex et le risque de migration précipité sur les territoires de l'Union en 2021. Les tensions avec la Biélorussie ont provoqué ce qu'il faut appeler une crise frontalière résulter d'un afflux massif de migrants du Moyen-Orient au nord de l'Europe en 2022, c'est évidemment le conflit en Ukraine qui a conduit à des déplacements de populations entières vers les territoires des États, dans dans certains cas il ne s'agit aucunement de crise migratoire au sens strict de mouvements de population spontané, ni même de simples questions d'asile et de droits de l'homme. Il s'agit de tentative de déstabilisation étrangères et de péril pour notre sécurité commune. Or plus importants sont les flux migratoires plus importants sont ces défis sécuritaires plus forte doit être la réponse de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle Frontex constitue désormais outre un moyen de coordination de nos frontières. Une force opérationnelle qui doit être capable de se projeter dans ces zones afin de soutenir les États concernés. L'échelle continentale de nos frontières. Et l'ampleur des flux migratoires l'exige. En 2ème lieu, la finalité de l'action de Frontex est resté inchangé c'est de préserver l'ordre et la sécurité jusqu'aux frontières extérieures de l'Union européenne. Or là encore les défis se sont multipliées durant ces dernières années, accroissant les missions confiées à cette agence. C'est d'abord le cas en raison du terrorisme international qui doit qui rend nécessaire une maîtrise accrue de nos frontières et une plus grande vigilance à l'endroit des zones de conflit. C'est également le cas de la criminalité transfrontalière elle aussi venues s'ajouter aux missions de Frontex depuis 2016. C'est enfin le. Il des trafics se déroulant dans les zones frontalières et nécessitant un appui des États membres. Il en résulte de nouveau un accroissement salutaire des moyens et des capacités opérationnelles de Frontex puisque l'agence est appelé à intervenir au soutien des États et parfois directement sur le terrain. Un constat d'ensemble s'impose ainsi à tous les États membres et à l'Union elles-mêmes. Nos frontières ne peuvent se réduire à de simples zone d'accueil, nos États ne peuvent faire face seuls aux défis géopolitiques et sécuritaires du continent tout entier. L'élargissement du mandat de Frontex et la croissance de ses moyens opérationnels sont d'une évidente nécessité. C'est ce qui doit conduire cette organisation à devenir la plus large agence européenne tourné vers le maintien de l'ordre. À nos frontières et la bonne application de notre politique migratoire. Nous voudrions insister sur la croissance naturelle de cette agence qui justifie pleinement l'adoption sans modification de cette proposition de résolution par la commission des affaires européennes, elle n'est pas seulement naturel parce qu'elle répond aux défis que nous venons de souligner. Elle est également logique car elle s'inscrit dans le prolongement de nos propres valeurs républicaines en 1974 Raymond Barre déjà lors d'un discours de politique générale l'importance d'élargir notre attention envers la liberté, la responsabilité, la sécurité, la raison d'être de Frontex ne s'en écarte pas le contrôle des frontières extérieures contre l'immigration irrégulière contre les pressions étrangères contre l'insécurité dans l'Union européenne. Ne laissons pas croire que la liberté implique l'insécurité c'est tout au contraire la sécurité que nécessite la liberté. La proposition de résolution de nos collègues, Jean-François Rapin et François Noël Buffet il répond pleinement en soutenant l'agence Frontex. Elle vise à la stabiliser efficacement au plan politique et juridique. Juridiquement il faut acter l'irréversibilité du mandat accordé à Frontex. Il s'est accrue en 2016 et ses moyens opérationnels doivent accompagner cette croissance. L'enjeu de sécurité frontalière s'en trouve satisfait d'une part Frontex nerfs bien n'intervient qu'à la demande des États. Il ne revient pas à l'agence de les surveiller, ni même d'intervenir par elles-mêmes mais de les soutenir. Quant au maintien de l'ordre à leurs frontières. D'autre part la coordination de la lutte contre la criminalité transfrontalière l'immigration irrégulière et la sécurité intérieure s'avère préserver dans les strictes conditions déterminées par les États. Il faut également appuyé au plan politique. L'autorité de son futur directeur exécutif. La place institutionnelle de Frontex au sein de l'Union européenne et la crédibilité internationale de cette dernière s'avère lié par cette condition C'est pourquoi nous voudrions réaffirmer ici tout le soutien que nous apportons à Frontex, y compris et jusqu'aux critiques et aux polémiques dans cette agence a fait l'objet. Accordons-nous, chers collègues, sur au moins un point à cet égard. Quelles sont les conclusions des rapports consacrés à l'activité de Frontex par ailleurs cité dans les travaux préparatoires de cette proposition de résolution si Frontex n'a pas participé directement à des opérations de refoulement. Il ne les a pas empêchés. Si les incidents et les atteintes aux droits fondamentaux ont révélé des insuffisances structurelles dans leur traitement et si les cadres dirigeants se sont plaints de l'ignorance des enjeux opérationnels de l'agence. Que manque-t-il à Frontex. Si ce n'est davantage de moyens précisément afin de pouvoir garantir le respect des droits fondamentaux. La seule introduction en 2019 d'un officier aux droits fondamentaux, assisté de contrôleurs et d'un code de conduite ne suffit pas. pour que ces garanties devienne effective jusqu'au coeur des missions opérationnelles de Frontex. Il faut continuer à les soutenir et à lui fournir les moyens nécessaires les recommandations jointe à cette proposition de résolution convergent utilement avec cette croissance de moyen accroissement de la transparence. Instauration d'un contrôle parlementaire. Soutenir Frontex ainsi que surmonter sa crise de croissance et sa crise de confiance ne se ne peut s'accomplir qu'en augmentant ses moyens. Et, d'une part en lui exprimant notre assentiment. D'autre part, je vous remercie. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues d'ici quelques semaines, nous examinerons le projet de loi visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, la gestion des flux migratoires, l'un des sujets majeurs de nos politiques publiques de ces dernières années et les controverses récentes autour de l'agence Frontex. Non, certainement pas participer à apaiser le débat. Au point de le relancer. Quant au sens de la mission de Frontex. Chacun le sait ici, il y en a 2 principales et pour reprendre les termes du règlement de 2016 instituant l'agence. La première est de faciliter et rendre plus efficace l'application de mesures de l'Union européenne. Relative à la gestion des frontières extérieures, la seconde de contribuer à l'application du droit de l'Union à toutes les frontières extérieures, notamment en matière de droits fondamentaux. Faut-il alors être gêné par cette seconde mission et ne retenir que la première l'une et l'autre ne paraissent pas de 5 compatibles à condition d'être menée sans dérive et avec la confiance réciproque de chacun des États. Ce qui devrait aller sans dire en Europe. Seulement nous touchons là au vrai problème que rencontre Frontex. Il ne tient pas simplement à des affaires de statut. Car ce ne sont pas quelques lignes dans un règlement qui donneront sa légitimité à une institution, ce sont les faits les décisions et les actes de ceux qui la font vivre et de ce point de vue, tout le monde est unanime pour souligner les manquements les dérives et les fautes commises ces dernières années. Je ne mets pencherait pas sur la démission de son ancien directeur exécutif en lien avec le rapport de l'Office de lutte antifraude européen ainsi que des accusations d'avoir couvert des opérations de refoulement de migrants vers la Turquie par la Grèce. Entre 2019 et 2020. Il en ressort une véritable fragilité pour l'agence, mais qui peut être une opportunité et un cap pour son nouveau directeur. Celui-ci semble en avoir conscience puisqu'il s'est engagé à rétablir la confiance dans l'agence, que beaucoup de nos concitoyens ont perdu. Et c'est là que se trouve le véritable enjeu de ces prochaines années pour Frontex. Il a été largement souligné par les orateurs précédents combien les moyens mis à disposition de Frontex était important. Celle-ci dispose en effet de moyens juridiques renforcée pour assister les États membres par exemple dans le suivi des flux migratoires. Le contrôle des frontières, la lutte contre l'immigration illégale et les réseaux criminels transfrontaliers mais également dans l'organisation des opérations de retour des migrants n'ayant pas le droit de rester sur le territoire de l'Union européenne. L'Agence devrait également être doté de moyens matériels et humains supplémentaires à savoir notamment un contingent permanent de 10.000 garde-frontières et garde-côtes à échéance 2027 ainsi qu'un avion qui est d'ores et déjà en action dans la Manche. Un tel dispositif ne peut être accompagnée d'autant de controverse, il nous faut oeuvrer à sa stabilité dans ces deux missions initiales qui vont de Pair. En revanche. Il y a un point sur lequel je rejoins davantage les auteurs de cette proposition de résolution celui du rôle des parlementaires nationaux. Vous proposez qu'ils soient mises en place dans chaque parlement national. Je cite un groupe de contrôle parlementaire sur le modèle de celui établi pour contrôler les activités d'Europol, afin de garantir la nécessaire association des Parlements nationaux au contrôle de Frontex. Si notre groupe rappelle régulièrement son attachement à la construction européenne et plaide pour que les institutions créées au niveau de l'Union affirment leur légitimité sans qu'il faille nécessairement les associer aux institutions nationales que face aux crises et lorsque nous sommes dans un processus de reconstruction d'une légitimité comme Frontex. Le rôle des Nations, être essentiel. Il permet d'observer et de réguler afin de pouvoir faire confiance à nouveau. Certes, l'agence est actuellement responsable devant le par l'Europe. Le Parlement européen et le Conseil mais je crois que cette idée d'un contrôle parlementaire au niveau national participera à justifier ses actions à l'avenir et à éviter de nouvelles crises. En conclusion, malgré certaines réserves. Nous comprenons RDSE les enjeux de cette proposition de résolution notre groupe se prononcera donc en faveur de celle-ci. Je vous remercie. Merci, chers collègues, la discussion générale est Close. Nous allons passer la discussion du texte de la proposition de résolution européenne. Qui a un article unique sur lequel j'appelle d'abord l'amendement numéro 4. Présenté par Monsieur Fernique et ses collègues. Monsieur le président. Chers collègues, la sécurisation de nos frontières doit passer par le rétablissement de l'espace Schengen. Suspendu, on le sait depuis 2015 et par une refonte totale de la politique d'accueil de l'Union européenne pour renforcer la solidarité entre ses États membres et favoriser un accueil digne des personnes exilées réfugiés. C'est l'objet de cet amendement. Quel David la commission. Monsieur le rapporteur. La la commission émet un avis. Défavorable et cet amendement ne lui semble pas opportun pour, pour 2 raisons. D'abord parce que bien évidemment. Contrôle des frontières et qualité de l'accueil ne sont pas incompatibles. Et il pourrait même estimé qu'au contraire préserver l'intégrité de l'espace Schengen permet de prémunir notre système d'accueil contre les risques de saturation. c'est donc ainsi oeuvrer pour une solidarité finalement plus active. Et puis l'amendement précise lui-même qu'il ne ne vaut que dans le cadre. Je cite d'un fonctionnement normal de l'espace Schengen. Je crois que nous ne pouvons partager. Chers collègues, que la situation actuelle ne ne relève pas d'un fonctionnement normal. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Ministre. Le président. Contrôle harmoniser efficace des frontières extérieures est effectivement le corollaire indispensable à la libre-circulation à l'intérieur de l'espace Schengen et ce depuis la création de cet espace. Une politique d'accueil fondé sur la solidarité est effectivement essentiel à l'échelon une européenne. C'est d'ailleurs le sens du pacte sur l'asile et la et la migration proposé par la Commission européenne. Fin 2020, actuellement en cours de négociation. avec le Parlement et qui doit justement permettre d'améliorer le cadre juridique européen de l'accueil et de la solidarité entre les États membres et que soutient la France Il fait référence dans une résolution relative à l'agence Frontex ne m'apparaît pas pertinent. Ça ne cette agence n'exerçant pas de compétence en la matière. Le gouvernement donne donc un avis défavorable à cet amendement. Y a-t-il des explications de vote, s'il y en a pas je mets aux voix cet amendement avec les deux avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. L'abstention. N'est pas adopté. Nous passons l'amendement cinq également proposé par messieurs Ferrandi qui a la parole. Monsieur le président. Chers collègues pour cet amendement. La France devrait plaider au Conseil pour une refonte structurelle et complète de l'agence en conformité avec le droit international l'asile en vigueur cette refonte devrait notamment s'appuyer sur la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et son principe de non-refoulement des personnes aux frontières. L'avis de la Commission maintenant. cet amendement transforme en fait Frontex en en organisme de exclusivement dédié au sauvetage en mer et au secours en mer, donc bien évidemment cela ne va pas dans le sens. De la proposition. Ni de la position de la de la commission. Je voudrais quand même en rebond au. au fait ou contrefaits qui sont présentés dans l'amendement. Rappelez. Rappelez 3 points. Tous les rapports et puis on rebond aussi à quelques interventions discussion générale, tous les rapports, y compris du Parlement européen ont conclu à l'absence d'un. de proactivité en push Back en refoulement de de de front de de Frontex et en absence de responsabilité. Devrait rappeler aussi que les 40 contrôleurs ont déjà été. Embauchés. Au, au moment où nous nous parlons. Dire que les mécanismes de contrôle internes ont été considérablement renforcer les mécanismes de réponse ont considérablement été renforcée sur préconisation de la médiatrice. Qui de l'Union européenne qui a qui Qui a explicitement dans son rapport, insisté sur ce point et donc. Voilà ces quelques faits rappeler. Je crois conforte l'avis défavorable qu'il m'incombait d'exprimer. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Monsieur le président. Bien évidemment le gouvernement est très attaché au respect du droit international. Du principe de non-refoulement. Et les droits fondamentaux des migrants. Toutefois, la refonte du règlement Frontex aujourd'hui nous paraît très prématuré, notamment dans la mesure où une évaluation de ce règlement est en cours. Elle n'est pas nécessaire aujourd'hui pour améliorer la protection des droits fondamentaux dans les actions de l'agence. Le règlement actuel telle qu'il ait. Prévoit en effet toutes les garanties nécessaires et c'est plutôt sur sa mise en oeuvre. faut se concentrer. Par ailleurs, les recommandations du groupe de contrôle du Parlement européen que vous proposez de soutenir sont déjà mises en oeuvre des 44 contrôleur des droits fondamentaux sont recrutés depuis fin 2022 le nouveau mécanisme de remonter des signalements des incidents. Notamment en cas de violation des droits fondamentaux a été adoptée le 19 avril 2021. Cela est déjà fait. En août, le gouvernement partage pleinement le sens de la révolte résolution sur ce point. L'enjeu pour Frontex et d'abord la mise en oeuvre pleine et entière de son mandat, 2019 dans un contexte géopolitique nouveau cette tâche est importante, il nous faut stabiliser le mandat de cette agence pour qu'elle exerce enfin pleinement, complètement et sereinement. Enfin des discussions sur les à d'opérations de recherche et de sauvetage de rôle des ONG sont en effet essentiel dans le contexte actuel, elles ont lieu au niveau européen dans le cadre d'un plan d'action qui fait suite à la réunion demandée par le ministère de l'Intérieur. Donc j'ai fait état toute à l'heure. Il me semble que cette question dépasse largement le compteur de l'agence Frontex. Il doit être traité avec toutes les parties prenantes et non pas simplement sur le règlement intérieur de Frontex. L'action se déroule par ailleurs au sein des instances européennes respectons cette action pour être plus efficace, avis défavorable. Je voulais essayer de comprendre par rapport à ce que vient de dire monsieur le monsieur rapporteur et Monsieur le le ministre-parce qu'en fait dans ce qu'ils viennent de dire est-ce qu'il viennent des Despé qui effectivement si la nomination des 40 officiers de protection sont déjà fait et sont déjà effectifs si la création d'un mécanisme efficace de de signalements existe déjà c'est bien justement l'objet de cette résolution et que c'est pour ça qu'il faut l'inscrire dans la résolution. Donc je comprends pas où est le blocage c'est bien le but d'avoir une résolution de de donner de clarifier les orientations de Frontex. Donc si en plus vous me dites que c'est déjà fait, tant mieux. Parfait. Il faut justement l'inscrire dans cette, dans cette résolution et l'autre aspect qui est la France portera les recommandations du groupe de contrôle de Frontex dans son rapport rendu le 21 juillet 2021. Ça me paraît aussi assez logique.

Je mets aux voix donc l'amendement. Numéro 5 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Contre.

compte tenu de ce que nous avons indiqué en discussion générale sur la nécessité d'une indépendance strict. De l'officier aux droits fondamentaux et des personnes qui travaillent avec lui, de proposer des corrections dans la rédaction de ces alinéas de manière à ce qu'ils puissent bénéficier d'une indépendance totale et non pas. Par exemple, avoir à. Rendre compte devant le conseil d'administration. Un conseil d'administration qui selon la résolution. Doit être responsable de l'évaluation professionnelle de ces personnes, ce qui est une atteinte à leur indépendance. C'est la raison pour laquelle nous proposons ces modifications de rédaction qui sont essentiels pour sortir Frontex de la crise qu'elle a vécu. Quelle est la position de la Commission monsieur le rapporteur. L'opposition et et. L'amendement est contraire à la position de la commission qui a trouvé. Un Un équilibre. Et nous souhaitons le concert. Oui. Monsieur le Ministre ne vis à vis du gouvernement. Parlement est favorable à cette proposition d'amendement à double titre, il est favorable à l'indépendance de l'officier des droits aux droits fondamentaux et des contrôleurs des droits fondamentaux. Cette garantie d'indépendance et d'ailleurs déjà prévue par le règlement de Frontex, qui dispose que ceux-ci agissent en toute autonomie et en toute indépendance et dispose des ressources humaines et financières nécessaires. Le gouvernement n'estime donc pas nécessaire que le gouvernement que le conseil d'administration de Frontex propos procède à l'évaluation professionnel de ce dernier, ce qui serait difficile à concilier avec les garanties d'indépendance que la loi européenne prévoit. Cela n'exclut pas que l'officier chargé des droits fondamentaux rendent compte au conseil d'administration et la France, il est attentif. Elle a par ailleurs candidaté pour représenter le conseil d'administration dans un groupe de travail relatif à l'exercice de la mission de l'officier aux droits fondamentaux. Par ailleurs et plus fortement. Monsieur le rapporteur. Si l'expérience de gardes frontières peut être une ressource professionnelle utile pour l'exercice de la mission d'officiers de contrôle de droits fondamentaux, ce ne peut être une condition préalable d'autres compétences peuvent être qui la maîtrise des procédures, la maîtrise du droit international humanitaire, le sens des situations ainsi qu'une certaine culture géopolitique. En outre, et c'est peut-être le plus fondamental. Grimm Eden est déjà nommé actuel officier chargé des droits fondamentaux. Il a pris ses fonctions en juin 21 émettre une telle recommandation. Aujourd'hui nous semble jeter le doute sur sa légitimité. Alors qu'elle a au contraire besoin d'être conforté la sienne comme celle des 45 contre l'un des droits fondamentaux déjà recruté par l'nous souhaitons. Le nous soutenons donc cet amendement.

Une bonne formation et une évaluation sérieuse de l'agent lui permet une certaine indépendance. Ce serait le fait de ne pas le former correctement et de ne pas comprendre le métier des autres avec qui il va travailler en permanence qui serait un rejet de son indépendance. je crois que c'est important de savoir. Comment exercent leur métier. Vous dites Y a-t-il d'autres explications de vote non. Alors sur ce. Sur cet amendement, je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains et donc nous allons l'annoncer. Il va être procédé au scrutin dans les conditions de l'article 56. Ça Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Donc, le scrutin est clos. Nous allons voir le résultat.

Monsieur le président. Dans la même. Dans la même veine que le précédent. Nous considérons qu'il n'est pas acceptable de laisser la rédaction de le de La Linea 45 sous la forme rappelle que l'émission de Frontex et en aucun cas de surveiller les actions des États membres en matière de droits fondamentaux. Nous considérons au contraire que la crédibilité de Frontex dans ses actions et de veiller au respect des droits fondamentaux dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle nous proposons des modifications de rédaction à cet alinéa. Entendu. Quelle est l'opinion de la commission. Monsieur le rapporteur. monsieur le président. La première partie de cet amendement proposé par le groupe socialiste précise que la mission première. De Frontex n'est pas de surveiller le respect des droits fondamentaux par les États. Nous avons là un désaccord cas ce n'est pas une question de de hiérarchie. La mission de Frontex n'est tout simplement pas de surveiller les États, ni à titre principal, ni à titre accessoire. Comment les États pourrait-il solliciter son intervention. Quoi qu'il en soit, l'article 10 de du mandat de Frontex est très clair sur ce point tout cela n'enlève rien au fait que l'agence doit elle-même agir dans le respect des droits fondamentaux et que ces agents doivent signaler des manquements dont ils seraient témoins au titre de l'article 46 de son mandat. Frontex peut même aller jusqu'à se désengager d'une opération conjointe. la Commission avait néanmoins émis un avis favorable sous réserve de la suppression de la première partie de l'amendement. Car nous nous retrouvons sur la seconde. Celle-ci. Paraît apporter un complément intéressant une précision intéressante à la paix, Pierre et l'auteur de l'amendement. Ah je crois. Mais peut-être a-t-il changé de point de vue souhaitez le maintenir. En l'état, auquel cas je serais navré de devoir émettre un avis défavorable sur l'ensemble de l'amendement. Monsieur le ministre, le gouvernement partage totalement l'avis de monsieur le rapporteur. Et dans ses contradictions, si le l'amendement n'est pas modifié. Il s'en remettra à la sagesse. Du Sénat. Monsieur le comte sur cette suggestion de modification d'amendements. Quelle est votre réponse. Écoutez. Je veux bien modifier l'amendement finalement ça ne changera pas notre vote final mais s'améliorera malgré tout la rédaction de la pépère. Même si je regrette que ce ne soit pas l'ensemble de l'amendement parce que finalement cet amendement, il est au coeur de la crise. Parce que Frontex doit pouvoir témoigner de tous les manquements aux droits fondamentaux dont ils sont témoins. C'est la raison pour laquelle c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait. Qu'ils ont été que que nous avons vécu cette crise. Voilà maintenant j'accepte de de de de de de maintenir sa planque le deuxième partie de l'amendement de manière à ce qu'il puisse être adopté et participer à une amélioration de la pépère voilà merci. Ça fait disparaître le grand hein sur le document que nous avons sous les yeux et donc sur le l'amendement rectifié qui serait le grand de nous constatons à la vitre du coup favorable de la commission et toujours un avis de sagesse du gouvernement.

Monsieur le comte à nouveau l'amendement numéro 3.

de de de de de l'État avec lequel les opérations conjointes sont menées. Toutefois, nous estimons qu'il n'est pas raisonnable de mettre dans cette pépère le la phrase estime que les personnels de Frontex ne saurait être tenue juridiquement responsable d'éventuelles actions litigieuses commises dans le cadre d'opérations conjointes par les services de l'État partenaire. N'ont rien si si les personnels de Frontex n'ont rien fait ils n'ont pas à être. Responsable juridiquement. Toutefois, nous ne pouvons pas proposé d'immunité au personnel de Frontex. Quoi qu'il arrive, dès lors que ce sont des opérations conjointes donc c'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet amendement.

il ne s'agit. Il s'agit uniquement. De bien dissocier les responsabilités de chacun. Et de et de plaider par cet alinéa pour que la responsabilité des agents de Frontex ne puisse être engagée pour d'éventuels manquements aux droits fondamentaux commis par d'autres. ça me paraît être la du bon sens mais malheureusement. Rendue nécessaire. Dans l'écriture est rendue nécessaire par les par les faits et les accusations parfois portées à tort. Ces derniers temps. ils ne sont pas immunisés contre des poursuites pour des faits dont il serait directement les auteurs. Cela va mieux en le disant mais soit tu mais il n'y a rien d'écrit contre et l'article 86 du règlement de de Frontex et et plus qu'explicite sur ce point. Ils sont traités de la même façon que les agents de l'État hôte. C'est clair. Et puis enfin. Les agents ne sont pas et que ce n'avait non plus de reporter des incidents dont ils seraient les témoins. Via la procédure de signalement des incidents graves qui, je le rappelais tout à l'heure a encore été améliorée et conforter. Que l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Des agents de l'Union européenne, il n'est pas, me semble-t-il. Question d'immunité absolue des personnels de frontière. Ces derniers doivent en effet pas tenu responsable lors il n'a aucun contrôle. Sur les actions commises par les services de l'État hôte en revanche les personnels de Frontex sont tenus à un strict code de conduite applicable à toutes les personnes. Participant aux activités de l'agence, ils doivent garantir la protection des droits fondamentaux des personnes dans toutes leurs activités et ils sont à cet égard déjà tenus de signaler tout incident ayant potentiellement violé les droits fondamentaux des personnes au cours d'une opération de l'agence le responsabilité s'étend donc et c'est ce que je veux souligner particulièrement au signalement d'action litigieuse. Elle peut être engagée sur ce terrain. En revanche la responsabilité directe pour les faits litigieux commis par des services de l'État partenaire sur lesquels ils n'ont pas de contrôle n'est pas engagé. Il me semble donc que le texte de la résolution. Et tout à fait compatibles avec la réalité opérationnelle il n'invite pas pas du tout institué un régime d'immunité et c'est donc pour ces raisons que le gouvernement est défavorable à l'amendement proposé. Il y a donc 2 avis défavorables, y a-t-il une explication de vote n'pas donc je mets aux voix. Cet amendement numéro 3 double avis défavorable qui est pour.

les signalements ne sont pas faits. Je crois que nous pouvons retirer cet amendement. Ça permet d'atténuer finalement la rédaction de de la pépère qui. Peut donner cette impression. Merci. Il nous reste un amendement numéro 6 de monsieur Fernandes, qui va le défendre. Frontex. On l'a dit et l'agence la plus dotée de l'Union européenne, pourtant elle pose problème au regard du droit international et européen comme l'a révélé l'enquête de l'Olaf. Les millions d'argent public investi. Qui finance cette agence devraient donc servir à financer une vraie politique de contrôle et d'accueil qui soit compatible avec les valeurs fondatrices de l'Union, c'est le sens de cet amendement. La position de la Commission sur cet amendement numéro 6 monsieur le rapporteur. le rôle et les missions. À Frontex que la commission veut voir conforté et cette proposition aussi. Sont totalement antagonistes de l'approche.

Il me semble que la plupart des propositions présentées dans cet amendement sont déjà prévues. Dans le droit de l'Union européenne applicable aux frontières extérieures. Information des migrants Access. Juridique, enregistrement des demandes d'asile prise en compte des vulnérabilités ou font l'objet en ce moment. De négociation dans le cas du pacte européen sur l'asile et l'immigration par la Commission européenne fin 2020.

ne relève pas du mandat de l'agence Frontex inquiets seulement. Sur les frontières extérieures et la rédaction de cet amendement laisse à penser que les choses sont un peu mélangé entre les frontières extérieures les frontières intérieures,

antagonique avec le sens et les missions de Frontex et pour l'autre. Notre amendement. Liste. Des missions des des des, toute une série de choses qui sont déjà assurés dans le fonctionnement Frontex. J'avoue ma perplexité. Il faut quand même voter. S'il y a pas d'autres, d'explication de vote donc je mets aux voix cet amendement numéro 6 avec avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Contre. L'abstention. Merci. Donc il n'est pas adopté et nous concluons avec l'amendement numéro 7 également présenté par notre collègue Fernie qui qui a la parole. leur permet de fait d'échapper à leur obligation internationale en toute impunité. La sous-traitance notamment entraîne des atteintes forte au respect des droits fondamentaux qui se sont aggravées ces 5 dernières années on le sait. Face à l'échec du règlement de Dublin. La France devrait promouvoir au Conseil une politique d'accueil et de contrôle plus intégrée et solidaire et plus généralement un régime commun de l'asile européen, c'est ce que propose cet amendement. Et la position de la commission. Monsieur le rapporteur. Et défavorable. Le ministre. Le gouvernement entend tous ces arguments et il n'est pas favorable à l'externalisation Rwanda ou je ne sais où, de, de, de choses comme ça mais je pense que c'est un amendement politique qui est respectable mais qui n'a pas sa place dans cette résolution, avis défavorable. Donc. À d'autres demandes d'explications de vote, donc de la commission et le gouvernement donne de la ville est favorable je mets aux voix qui est pour. Qui est contre. Abstention n'est pas adopté. Je dois donc maintenant mettre aux voix l'ensemble de la proposition de résolution donc son article et les les les termes précédent le l'article unique et. Y a-t-il des demandes d'explications de vote sachant que nous allons avoir un scrutin public. Monsieur le Président buffet. Merci monsieur. Juste un mot. Pour indiquer que cette résolution. Elle a pour but aussi de marquer la nécessité d'un équilibre. Nous avons en réalité aux problème de migration. De loi qui s'applique une loi nationale est évidemment une réglementation européenne, les deux ne peuvent pas être. Antinomique et nécessairement. Nous avons besoin de cet équilibre. On a bien noté la volonté du gouvernement de renforcer sa politique migratoire. On en débattra dans quelques semaines et il est important aussi, qu'à l'échelle européenne les moyens soient donnés pour que la protection des frontières extérieures de l'Europe soient protégés. C'est le seul point que je voulais soulever tout en redisant aux collègues que naturellement pour nous. Il n'est pas question que les droits fondamentaux de ce qui arrive ne soit pas respectée et que tout l'enjeu de Frontex aujourd'hui c'est de retrouver une organisation sincèrement sincèrement apaisé. On peut le dire très clairement et puis qui se retrouvent dans sa mission première mais qui naturellement se soucieuse des droits fondamentaux des uns et des autres, je dois dire que.

de difficultés particulières, en tous les cas, pas celle qu'on a pu imaginer en Grèce. Plus récemment mais qui néanmoins il faut quand même faire confiance à l'institution dans son organisation aujourd'hui pour remplir correctement sa mission. Merci. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre. Nous voterons contre cette proposition de résolution européenne car nous considérons que. Elle ne marque pas suffisamment l'indépendance des contrôleurs des droits fondamentaux, sortir et des qui aurait permis d'éviter la crise que Frontex a connu. Parce qu'il y a une difficulté systémique. Que j'ai indiqué lors de la discussion générale ce que Frontex n'intervient que sous la responsabilité des États membres. Et que par conséquent. Il y a quand même une difficulté si on considère que pour le bien des frontières de l'Union européenne, il faut effectivement Frontex accompagne un État-membre mais que Frontex constate des dysfonctionnements. De de de l'État membre considéré et ne peut pas les dénoncer parce que sinon voilà il y aura plus de vrai. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est absolument indispensable qu'une indépendance totale, c'était la raison de notre premier amendement. Ça n'a pas été suivi. Donc nous considérons que nous n'avons cette proposition de résolution ne permet pas de tracer des pistes qui sortent Frontex d'une situation de crise, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette résolution. Merci. Maintenant le président lapin. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre quelques instants pour abonder bien sûr les les propos du du président buffet et avant de passer au vote. Je pense que la parole de chacun s'est exprimé. Et chacun dans sa diversité et de façon de façon correcte et, et je vous en remercie tous. Cette proposition de résolution avait été adoptée en en commission des affaires européennes. Si ce soir le vote là confirme. Le gouvernement j'espère on tiendra compte. Mais c'est pour vous dire aussi que plus que jamais et je pense que les événements. Des des dernières heures doivent nous inciter à une certaine vigilance aussi sur les La question migratoire qui va se produire suite au séisme et c'est Patricia Schillinger qui gentiment est venu nous. Nous dire mais que va-t-il se passer. Dès lors que ce séisme en en Syrie en Turquie, qui a fait de nombreux morts mais aussi pour d'autres raisons de nombreux gens à la rue risque de prouver de de provoquer un afflux migratoire conséquent et plus que jamais, nous aurons besoin des agents de Frontex. Moi je les ai vus travailler, je ne suis ni un procureur ni un distributeur de bons points mais tout ce que j'ai vu ce sont des gens qui travaillés. Comment. un c'est un. Je ne vous ai pas coupé Madame Benbassa quand vous avez parlé. Et donc je je pense que voilà, nous aurons plus que jamais besoin d'une agence Frontex forte avec des gens responsables respectueux des droits fondamentaux et je pense qu'elle a pris des dispositions. Avec la nomination des agents des gardes des agents et des gardes. Pour surveiller les frontières, à la fois pour garder les frontières mais aussi pour respecter justement ces droits fondamentaux. Entendu donc n'est plus de demandes d'explications de vote et je mets aux voix l'ensemble de la proposition. Et nous avons été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains, il va être procédé au scrutin dans les conditions du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est donc clos. Et. Voilà. Nous pouvons annoncer le résultat votants 344 exprimé également 344 pour la résolution 252 voix et contre 92 la résolution donc adopté. En application de l'article 73 qui acquiesce 4ème alinéa du règlement. La résolution que le Sénat vient d'adopter sera transmise au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Chers collègues, je vais levée prochaine séance jeudi, demain à 10h 30 pour les questions orales. La séance est levée.